La séance est ouverte, le compte rendu intégral de la séance du mercredi 11 octobre a été publié sur le site internet du Sénat : il n'y a pas d'observation. Le procès verbal est adopté. Conformément aux articles 56 et 13 de la Constitution, monsieur le président du Sénat, a saisi la commission des lois pour qu'elle procède à l'audition émette un avis sur la nomination de Madame Dominique Lottin qu'il envisage de nommer aux fonctions de membre du Conseil constitutionnel en remplacement de Madame Nicole Belloubet acte donner de cette communication. J'informe le Sénat qu'une candidature pour siéger au sein de la commission des affaires européennes a été publié cette candidature sera ratifié si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement. Par lettre en date du 12 octobre 2017 Monsieur Hervé Marseille, président du groupe Union centriste a demandé l'inscription dans son espace réservé du jeudi 26 octobre d'un débat sur le thème : Logement social sur quel territoire, comment et pour qui, demain, ce ce débat sera inscrit au sein de cet espace réservé avant l'examen de la proposition de loi tendant à simplifier certaines obligations applicables aux collectivités territoriales dans le domaine du service public d'eau potable, le président d'union du groupe Union centriste a également demandé que la durée de la discussion générale sur cette proposition de loi soit réduite d'une heure à 30 minutes il n'y a pas d'observation. Il en est ainsi décidé. Par lettre en date de ce jour, monsieur Claude Malhuret, président du groupe République et Territoires, les indépendants, a demandé l'inscription de 2 débats dans l'espace réservé à son groupe du mercredi 25 octobre sur les thèmes suivants l'Intelligence artificielle, enjeu économique et cadres légaux, la participation dans l'entreprise, outil de croissance et perspectives les débats inscrits dans ces espaces réservés pourrait être organisée sous la forme de questions-réponses, selon le principe retenu par la conférence des présidents réunis le 5 octobre dernier l'organisation proposée par la conférence des présidents pourraient faire l'objet d'un ajustement, le nombre de questions passerait de 17 à 21 avec la répartition suivante les républicains ces questions, le groupe socialiste républicain 4 questions, le groupe Union centriste 3 questions : la République en marche, 2 questions Rassemblement démocratique et social européen, 2 questions communistes, républicains, citoyens écologistes 2 questions, République et Territoires, les indépendants, une question : les non-inscrits, une question si les non-inscrits inutilisés pas leurs questions, elle serait attribuée au groupe les républicains, il n'y a pas d'observation. Il en est ainsi décidé, enfin, le Sénat ne siégera pas le soir du mercredi 31 octobre il n'y a pas d'observation, il en est ainsi décidé. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats du régime général et et de la prof des obligations. Dans la discussion générale, l'étape, la parole est à madame Nicole Belloubet Garde des Sceaux ministre de la justice.

d'un droit des obligations moderniser accessible et attractif, le gouvernement vous propose donc aujourd'hui de ratifier explicitement ce texte comme l'engagement en en avait été pris en 2015, alors même que votre assemblée avait exprimé clairement et fermement son opposition au principe de l'habilitation je ne reviendrai pas sur ce débat qui est maintenant derrière nous, je crois en effet qu'au-delà des questions de méthodes chacun ici s'accordera pour affirmer que cette réforme historique, entré en vigueur depuis un an maintenant, était devenu à la fois urgentes et indispensables. En effet, alors que des pans entiers de notre code civil avait été rénové au cours des décennies précédentes et je pense ici notamment au domaine du droit de la famille que des pays qui pourtant autrefois s'était inspirée du code Napoléon, c'était depuis affranchi de ce modèle, qui était jugé trop anciens pour demeurer, source d'inspiration et ces pays n'avait pas attendu pour réformer leur propre droit des obligations, le droit français des obligations était lui toujours régi par des dispositions inchangé depuis 1804. Depuis ce constat qui avaient été formulées à l'occasion du bicentenaire du Code civil en 2004, donc ni le principe ni le urgence de la réforme n'avait été remise en cause, pourtant, rien n'avait été fait, aucun processus législatif n'avait été enclenché l'habilitation accordé au gouvernement en 2015, a permis de mener cette réforme, dans des conditions de travail tout à fait exemplaire et de publicité que je voudrais aujourd'hui rappeler devant vous, l'avant-projet d'ordonnance a été transmis au président de la commission des lois de chaque assemblée au moment du débat de 2015, ce texte s'appuyait alors sur des travaux qui étaient menés sous l'égide des professeurs Catala éthérée, entre 2005 et 2011 donc ils avaient travaillé pendant plus de 5 ans sur ces sujets, ces projets doctrinaux, c'était d'ailleurs enrichi des apports des professionnels du droit, il m'mais aussi des acteurs économiques dès le vote de l'habilitation acquis en 2015, la chancellerie a rendu public un projet d'ordonnance qui a alors été soumis à une très vaste consultation publique consultation publique, d'une part sur le site internet du ministère et d'autre part adressé directement aux administrations concernées aux représentants des professions du droit des milieux économiques et également aux universitaires. Cette large consultation qui a été ouverte pendant plus de 2 mois, a permis de recueillir près de 300 contributions qui ont représenté plus de 3200 pages émanant d'universitaires de praticiens de représentants des entreprises, chacune de ces pages a été lue et analysée par la Direction des affaires civiles et du sceau que je remercie ici du travail qu'elle a effectué de très nombreuses réunions de travail ont été organisées avec l'ensemble des parties intéressées afin de leur souverain de leur soumettre les modifications envisagées à la suite de cette consultation publique. L'ordonnance qui a donc il était publié le 10 février 2016 n'est ainsi pas une oeuvre élaborés dans le secret d'un bureau ministériel, ce qui n'aurait pas été acceptable d'ailleurs, mais il est bien le résultat d'un travail fructueux et d'une collaboration hein. le seul examen comparé de l'avant-projet d'ordonnance et de l'ordonnance qui a finalement été publié, révèle la tension qui a été porté par le gouvernement aux critiques et aux propositions qui ont été formulées dans le cadre de cette consultation. De nombreuses améliorations ont en effet été apportées au texte, à la suite de cette consultation des améliorations, dont certaines étaient d'ordre technique, d'autres en réponse à des inquiétudes légitimes manifesté notamment par les acteurs économiques, c'est ainsi que le Champ d'application de la prohibition des clauses abusives a été restreint au contrat d'adhésion aucun critère tenant à l'Avantage manifestement excessif a été ajouté à la définition de l'abus de dépendance ou encore que le mécanisme de la sub-rogations conventionnel a été réintroduit. La publication de l'ordonnance sur le droit des contrats a part ailleurs été accompagnée de la publication d'un rapport de présentation au président de la République particulièrement substantiels puisqu'il fait plus de 50 pages ce rapport constitue pour le juge, comme pour la doctrine un remarquable outil pour les éclairer sur les intentions du gouvernement lors de l'élaboration de l'ordonnance ce rapport forme depuis l'entrée en vigueur de ce texte, un guide précieux pour les praticiens. Il aura ainsi fallu mesdames et messieurs les sénateurs, attendre près de 12 années entre le lancement des travaux à l'occasion des cérémonies du bicentenaire du Code civil et la publication de l'ordonnance du 10 février 2016 ces 12 années ont été particulièrement riche, comme je viens de vous le rappeler de contributions académique de réflexion d'échanges nourris entre l'ensemble des acteurs économiques, les professionnels du droit, et tout cela a entraîné de multiples consultations par l'ordonnance qui est entré en vigueur le 1er octobre 2016 ne constitue donc pas une révolution puisqu'elle est le fruit d'un travail construite progressivement et collectivement travail incessant de collaboration avec les praticiens qui ont tous eu à tous les stades de l'élaboration du texte, l'oreille attentive de la chancellerie, cette méthode de concertation qui a été salué par tous, a permis de mener à bien cette réforme dans le respect du double objectif fixé par la loi d'habilitation satisfaire à l'objectif constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, tout d'abord, mais également rendre le droit plus efficace et plus attractif, sans sacrifier l'intérêt des parties les plus faibles. L'ordonnance consiste avant tout et c'est le 1er objectif en une heure de codification de la jurisprudence remarquables abondante qui s'était développée depuis 2 siècles pour combler les silences du code civil ou adapter un texte devenu trop anciens, aux exigences de notre société contemporaine par essence fluctuante et donc source d'insécurité juridique, ces solutions jurisprudentielles largement admise, ont donc été inscrite dans le code civil pour plus de président prévisibilité par le texte de l'ordonnance. L'accessibilité du droit civil a également été renforcée par l'adoption d'un plan plus clair par un vocabulaire rénovés par des formulations plus simples, sans sacrifier à la tradition très française de concision et de clarté du code civil indispensables à sa pérennité. Le 2ème objectif, je vous l'ai dit, était le renforcement de l'efficacité de l'attractivité du droit français, en effet, ce droit des contrats rénover réaffirmera en tout cas, il est permis d'espérer la capacité de la France à servir de modèle en la matière. Les parties aux contrats internationaux qui peuvent choisir la loi applicable à leur relations pourront désormais pleinement s'en saisir, dans cette perspective, au-delà de l'abandon formel de la notion de cause, notion qui est incomprise de nos partenaires européens, notamment l'ordonnance consacre dans la loi, certains mécanismes issu de la pratique, telles que la cession de contrat ou la cession de dettes: l'ordonnance simplifie également d'autres dispositifs afin d'en rendre l'utilisation plus aisée, ainsi en est-il des formalités nécessaires à l'opposé, habilité de la cession de créances assoupli en réponse aux besoins de la pratique. Dans le souci de limiter le contentieux l'ordonnance développe les remèdes unilatéraux à la disposition du créancier, dans le cas d'une obligation in exécutés pour lui permettre de réagir rapidement en cas d'inexécution ces remèdes du sans avoir attendent l'issue d'un procès d'éviter une perte de temps et d'argent, qui peuvent être préjudiciable à la poursuite de son activité économique des solutions innovantes sont par ailleurs proposés à celui qui s'apprête à conclure un contrat ou à celui qui l'a déjà conclu à l'image des actions interrogatoire qui lui permettent de mettre fin à une situation d'incertitude juridique tels qu'un risque de nullité en mettant en demeure un tiers ou son co-contractant de prendre position sur cette situation dans un certain délai. Renforcer l'attractivité de notre droit n'impliquait pas pour autant de renoncer à nos valeurs traditionnelles et humaniste, le texte propose à cet égard des instruments garant de la justice contractuels protectrice de la partie faible tout en étant efficace et adaptée aux exigences de l'économie de marché. Au-delà de la consécration général du principe de bonne foi, l'ordonnance sanctionne ainsi l'exploitation abusive d'une situation de dépendance par un contractant ou les clauses, créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des partis, comme cela est déjà le cas dans les contrats de consommation notamment enfin est introduite la révision du contrat pour imprévision, ce qui permet l'adaptation du contrat, dont l'exécution est rendu excessivement difficile pour une des parties du fait d'un changement de circonstances indépendantes de la volonté des parties. Cette ordonnance, qui a intégré notre régime juridique depuis le 1er octobre 2016 et qui a nécessité un très important effort d'adaptation de la part des praticiens est aujourd'hui soumise pour ratification à votre assemblée. Si l'entrée en vigueur de l'ordonnance est encore trop récente, à peine un an pour permettre d'en apprécier en pratique l'incidence sur le contentieux : l'équilibre semble aujourd'hui être atteint entre la modernisation et le maintien des grands principes fondateurs de notre droit des contrats. Ainsi que la garde des Sceaux d'alors s'y était engagé devant votre haute assemblée, un projet de loi de ratification autonome a été déposé par le gouvernement et il est donc aujourd'hui inscrit à l'ordre du jour du Sénat cette ratification, mesdames et messieurs les et Naters impose,

socle des échanges économiques pour le simple particulier, comme pour la grande entreprise ou encore pour la très petite entreprise qui ne disposent pas de service. Mais Mais cette ratification était aussi un exercice qui suppose un grand esprit de responsabilité, comme l'affirmait très justement votre rapporteur, le sénateur François Pillet, le texte est en vigueur depuis le 1er octobre 2016 et il s'applique aux seuls contrats conclus depuis cette date, cette réforme, je vous l'ai dit a rendu nécessaire un important travail de mise en oeuvre, en particulier de la part des professions du droit et des entreprises qui ont dû adapter leurs pratiques, c'est pour prendre en compte ces considérations que le gouvernement avait d'ailleurs prévu une entrée différée des nouveaux textes au 1er octobre 2016. Il y a donc aujourd'hui un enjeu puissant en terme de stabilité de notre droit. Par des modifications substantielles du texte de l'ordonnance nous prendrions un risque : celui de créer un nouveau droit transitoire qui s'avère très néfastes en terme de lisibilité de sécurité juridique en renvoyant tu n'image d'instabilité, l'attractivité du droit français, pourtant poursuivi par la réforme s'en trouverait ainsi gravement compromise. Je souhaite à cet égard rendre hommage à l'état d'esprit qui a présidé au travail de votre commission des lois, et au travail de son rapporteur, Monsieur le Sénateur, en effet, le texte dont nous allons discuter démontre, si besoin était, que nous avons en partage, monsieur le rapporteur, l'impérieuse nécessité de préserver cette sécurité juridique sur certains points qui ne Vienne modifier ni le sens ni même l'esprit des textes, la commission a effectué des choix sur lesquels le gouvernement vous proposera tantôt de d'accepter, tantôt de revenir dans un seul but, celui de préserver l'ordre juridique établi depuis un an maintenant, et de ne pas créer, je me répète un nouveau droit transitoire la majeure partie des nombreuses observations qui ont été formulées par les commentateurs extrêmement nombreuses, qui ont écrit depuis la publication de l'ordonnance relève souvent de l'interprétation des textes à cet égard, je forme le voeu que les débats qui s'ouvrent maintenant sur cette réforme permet au gouvernement d'éclairer son intention et contribue à résoudre les éventuelles difficultés d'interprétation sans qu'il soit pour autant nécessaire de modifier substantiellement le texte pour conclure je nous convie collectivement à la prudence et à la prévoyance de Portalis qui, dans son discours de présentation du code civil nous mettait en garde et je le cite : il faut laisser le bien, si on est douteux : du mieux qu'en corrigeant un abus, il faut encore voir les dangers de la correction, même qu'il serait absurde de se livrer à des idées absolu de perfection dans des choses qui ne sont susceptibles d'une bonté relative qu'au lieu de changer les lois, il est presque toujours plus utile de présenter aux citoyens de nouveaux motifs de les aimer. Voilà ce qu'écrivait Portalis l'ordonnance qui porte, réforme du droit des contrats du régime général de la preuve des obligations et donc une étape historique dans l'adaptation de notre droit aux réalités du monde contemporain, quand bien même ce texte n'atteindrait pas aux yeux des plus sévère d'entre nous, un idéal de perfection, je vous invite, par les débats qui vont s'ouvrir à lui donner la valeur politique et symbolique que seule sa ratification peut lui conférer vous la ferait ainsi mieux connaître et qui s'est même peut-être mieux aimé de nos concitoyens, je vous remercie. La parole est à monsieur François Pillet, rapporteur de la commission des lois. Madame la présidente, madame la garde des Sceaux, le président de la commission des lois mais, chers collègues, le projet de loi de ratification que nous examinons cet après-midi, propose la ratification d'une ordonnance qui a réformé en profondeur, comme ça l'a été parfaitement dit par Madame la Garde des Sceaux, le droit des contrats, le régime général des obligations et le régime de la preuve des obligations, le Sénat s'était opposé à ce qu'il soit procéder par ordonnances certainement par principe mais beaucoup en l'espèce, parce que, comme l'avait souligné, notre collègue Thani Mohamed Soilihi, dans son rapport, s'agissant, je le cite, s'agissant de l'équilibre à retenir : entre l'impératif de justice dans le contrat qui peut justifier qui peut justifier une plus grande intervention du juge ou une modification des termes du contrat et celui qui s'attache à l'autonomie contractuelle et à la sécurité juridique du contrat qui peut justifier qu'une partie reste tenu par ses engagements même si lui deviennent défavorables, la réforme du droit des obligations pose des questions politiques majeures qu'il revient seul au seul Parlement de trancher, nous pensons encore et notre attitude restera la même, face à la pratique des lois d'habilitation même même si Madame Lagarde et vaisseaux dans le cas présent, le travail a indéniablement de qualité, le récit de l'imprévision la sanction des clauses abusives, le renforcement de lignes à terre à Nice où l'accroissement du rôle du juge, ce sont bien des choix politiques dont le Parlement a été privé au prétexte que cette réforme est essentiellement et faussement techniques, j'ajoute que le régime de l'imprévision va d'ailleurs au-delà me semble-t-il de ce qui figurait dans l'habilitation mais passons, nous nous accordions tous à penser que cette réforme était absolument nécessaire, il a fallu une décennie de réflexion françaises aiguillonné par des tentatives inabouties, l'harmonisation européenne, 2 piliers doctrinaux l'avant-projet Catala, l'avant-projet éthérée de multiples interprétations et construction jurisprudentielle un avant-projet de réforme publiés par le ministère de la justice en 2008 puis en 2000 11 heures consultations publiques en 2015, plus de 300 contributions adressées à la chancellerie et récemment, outre une gamme très large d'audition, une consultation par la commission des lois de l'ensemble des professions et juridictions des universités et des organismes intéressés pour restaurer un droit défraîchi. Et corriger une situation où le droit n'était plus dans le code, serait-ce quelques réserves, tenante en quelque sorte aux droits acquis en raison de l'application contrat antérieur des dispositions du code civil antérieur à l'ordonnance et à sa ratification, le Conseil constitutionnel nous laisse la possibilité d'exercer l'intégralité de nos pouvoirs de législateur, mais parce que c'est une réforme attendue globalement est largement approuvé le Sénat ratifiera. Parce que nous sommes en présence d'une ordonnance entrée en application et qu'il serait irresponsable dans l'histoire de l'évolution de nos règles juridiques de créer pour une période d'un peu plus de 12 mois. Une granule de droit mort-né, le Sénat ne proposera pas la réforme de la réforme, nous avons accepté de respecter les grands choix réalisés par l'ordonnance par exemple la suppression de la cause il ratifiera donc en poursuivant les 2 objectifs du gouvernement renforcé d'une part la sécurité juridique du droit des contrats en améliorant sa lisibilité, accessibilité et en renforçant d'autre part la tri l'attractivité du droit français, du point de vue strictement économique vis-à-vis des entreprises, mais également du point de vue de l'influence du système juridique français à l'étranger, le 1er de ces objectifs est essentielle à nos yeux, car l'latin du 2ème est impossible à vérifier dans l'attractivité du droit ne semble pas dépendre de facteurs étroitement juridique, une entreprise choisissant rarement un droit en fonction uniquement de sa qualité intrinsèque reste en 1er lieu certaines incertitudes sur l'interprétation qui pourrait être faite de dispositions qui, sur le fond ne suscite pas de critiques fortes et dire reste également des doutes sur la portée de règles contenues dans la réforme reste enfin des corrections nécessaires pour une plus parfaite cohésion nos qualifications juridiques et des pouvoirs dévolus aux juges dans notre droit des obligations et des contrats pour les premières or quelques affinement rédactionnel pour pas difficulté : la commission des lois proposées Sénat d'expliciter clairement et expressément l'interprétation qui doit être donné de textes qui pourrait éventuellement susciter des hésitations jurisprudentielles et d'incontournable loi interprétative le Sénat invite ainsi dans ces hypothèses particulière attachée au respect scrupuleux à ses travaux préparatoires qui sont source de droit, la commission des lois a validé toutes les interprétations qui figure dans mon rapport, j'invite les praticiens et les juges à s'y référer, par exemple, nous affirmons clairement que l'article 171 sur les clauses abusives ne peut pas s'appliquer dans les champs déjà couverts par le droit de la consommation, le droit des pratiques commerciales restrictives. Pour les seconds, concernant par exemple la capacité des personnes physiques ou morales ou l'application de la loi dans le temps les amendements retenus par la commission des lois qui ont été incorporées dans le texte soumis ce jour à vos débats, apporte des précisions nécessaires sans bouleverser l'objectif du texte ou sur l'architecture pour les derniers, je veux bien admettre que la discussion puisse être un peu plus ample, car il s'agit par exemple de définir avec précision : contrat de gré à gré et le contrat d'adhésion afin d'éviter des incertitudes, voire des contradictions qui ont été quasiment unanimement soulevées lors des auditions auxquelles j'ai procédé, il s'agit, par exemple dans cadrer les pouvoirs du juge face à des relations contractuelles bouleversé par un événement imprévisible qui avant octobre 2016 l'aurait pas été un moyen pour échapper aux obligations contractuelles ayant dicter la loi des parties sur tous ces points, nous verrons tout à l'heure au cours des des amendements, les débats qui pourront s'instaurer, mais Madame la garde des Sceaux au débat reste très ouvert, puisqu'il porte sur finalement peu de questions au regard des 300 articles concernés par la réforme, j'allais dire 10 questions mais il s'agit de points sur lesquels les critiques de la part des juristes professionnels les juges la doctrine sont quasiment unanimes : la commission des lois, on a tenu compte, pour parfaire une réforme dont je redis qu'elle a été bien menée, nous pouvons sans difficulté la parachever ensemble notons en conclusion pour nous en souvenir pour nous en souvenir que cette tâche aurait été définitivement plus aisée, s'il avait été définitivement renoncé à la mise en une application l'ordonnance avant leur ratification. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Pierre-Yves Collombat pour 6 minutes pour le groupe CRC. Madame la présidente, madame la garde des Sceaux, mes chers collègues, je ne saurais commencer mon propos sans saluer non seulement le travail approfondi mais l'effort de synthèse particulièrement éclairante de notre rapporteur sans rappeler non plus que nous continuons à penser que réformer le Code civil doit d'abord être l'affaire du Parlement avant d'être celle des fonctionnaires du ministère de la justice, aussi brillant et consciencieux soit-ils, ceci dit ce n'est pas principalement la procédure des ordonnances qui est critiquable en soi tous les correctifs sont en effet possibles au moment de la ratification, c'est leur mise en application avant ratification créant alors un droit spécifique à cette période de transition et bridant d'autant la liberté de manoeuvre du législateur législateur qui pour éviter cette complication supplémentaire avec raison en tient compte au moment de la ratification, il ne faudrait pas cependant que ces retards de ratification devienne un moyen de pression sur le Parlement, comment dit-on, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Ceci rappelé il y a, en l'espèce, notre groupe, considérant que ce texte atteint au moins 2 de ses objectifs : rendre le droit des obligations plus lisible et plus accessible en y intégrant une foisonnante jurisprudence renforcer la protection de la partie faibles, en introduisant la notion de bonne foi à toutes les étapes de la conclusion du contrat, celle de vice du consentement pour tenir compte de la violence de la vie économique, en corrigeant les éventuels déséquilibres entre les partis et en consacrant le devoir général d'information hé bien considérant tout cela, notre groupe ne voit aucune raison de s'opposer à cette révision quant au 3ème objectif : rendre notre droit plus attractif en adaptant le code civil aux besoins de l'activité économique affichage désormais obligatoire de la France aux Start-Up et me laisse rêveur d'abord parce qu'un droit qui devrait être attractif pour l'une des parties. Me semble-t-il le serait forcément au détriment de l'autre, le contraire du but de la réforme, ensuite parce que tout le monde, y compris des chefs d'entreprises anglo-saxon ne partage pas ce dédain pour notre propre droit. Mais est arrivé, en effet, de lire des témoignages de chefs d'entreprise anglo-saxon vantant la prévisibilité des décisions de notre pays, dans notre pays, par opposition des jugements dans notre pays, par opposition à leur caractère plus aléatoire dans le leur, nous approuvons aussi la plupart des modifications apportées par notre rapporteur au texte initial, à l'exception de quelques unes en nous sommes en désaccord avec la suppression du pouvoir de révision du contrat par le juge dans le cadre du nouveau régime de l'imprévision prévue à l'article 195 au motif qu'ainsi je cite le juge devient quasiment à un peu le 3ème partie au contrat nous semble jugement pour le moins excessif et surtout en contradiction avec l'esprit général de la révision qui est d'éviter, comme je l'ai dit les déséquilibres entre les parties en espèce le déséquilibre qui est créée par un changement imprévisible de la situation qui pénalise l'une seulement des partis il ne nous paraît pas non plus opportun de modifier la rédaction du 1er alinéa de l'article 233 je cite le créancier peu après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix formulation qui nous paraît plus souple, c'est la formulation initiale plus souple et tout aussi équitable que celle proposée par notre rapporteur enfin restreindre la notion de dépendance en la qualifiant d'économique ne nous paraît pas non plus un choix judicieux nous on la quasi Andy revenir donc lors de la discussion des amendements, amendements que donc c'est l'observation ont suscité réviser intelligemment le code civil, cependant, n'est qu'un préalable reste à appliquer cette révision qui suscitera inévitablement. Une période de flottement et donc probablement un surcroît de contentieux qui demandera que les juges civilistes dégage suffisamment de temps pour s'approprier toutes ces nouveautés, je ne ferai que reprendre les observations de l'USM, en conclusion de la note qu'elle consacre au présent projet de réforme, attirant une fois encore la tension, je cite, l'attention de la chancellerie sur le nombre inégalé de devoirs de vacance de postes de magistrats sur la surcharge généralisée des collègues sur l'impossibilité d'absorber à moyen constant des mots de nouvelles tâches et sur l'absolue nécessité d'inclure dans le calcul des États, des ETP le temps consacré à l'étude des modifications législatives, comment ne pas s'associer à ces propos. Je donne donc rendez-vous au gouvernement au projet doit une anse merci. Merci, cher collègue, la parole est à Madame Anne-Catherine Noisy pour le groupe UC pour 8 minutes. minutes. Présidente Madame Ministre, chers collègues, suite aux inquiétudes des chefs d'entreprise, la délégation aux entreprises du Sénat avait souhaité dès septembre 2016 être associés aux travaux de la commission des lois pour la ratification de cette ordonnance de février 2016 portant donc réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations, j'ai été chargé par la délégation d'examiner l'impact de cette ordonnance sur les entreprises, mais propos aujourd'hui qui seront donc ceux du groupe UC s'appuieront de fait très largement sur ces auditions auxquelles j'ai pu participer avec le rapporteur de la commission des lois, François Pilet, que je remercie pour son accueil et surtout pour le grand E intérêt l'enrichissement de ses entretiens. Quelques points de contexte a rappelé qui ont déjà été évoqués : tout d'abord, mais sur lesquels je pense qu'il faut insister tout d'abord le fait que cette réforme était largement attendu par l'ensemble des acteurs du droit mais aussi du monde économique dès 2006, la chambre de commerce et d'industrie de Paris souhaitait cette modernisation, je cite, à l'heure où le droit constitue non seulement un outil de régulation des échanges mais aussi un facteur de compétitivité économique en 2008 a déclaré à nouveau l'enjeu de la modernisation du droit des contrats ne se situe pas seulement sur le plan strictement juridique, mais s'appréhende également en termes de compétitivité de notre système juridique et d'attractivité de de notre territoire l'impact et les retombées attendues de cette réforme sont donc loin d'être négligeables et le rapport accompagnant l'ordonnance souligne fortement cette notion d'efficacité économique du droit 2ème point souligné qui a déjà été évoqué, c'est la marge effectivement limiter des pouvoirs du législateur pour modifier une ordonnance qui a, qui est de fait déjà entré en vigueur l'exercice des des donc pas simple pour pour notre rapporteur, puisqu'il s'agissait d'éviter une nouvelle source d'insécurité juridique un 3ème droit transitoire tant redoutée par les entreprises qui ne cesse de réclamer aujourd'hui une plus grande stabilité du droit

entre la modernisation du droit français et le maintien, vous l'avez dit, Madame la Ministre, de ces principes fondamentaux que sont la liberté contractuelle la force obligatoire du droit et son effet relatif, le Haut comité juridique de la place financière de Paris a rendu le 10 mai dernier un rapport rédigé sous la présidence de Monsieur Canivet qui soulignait encore cette contribution à l'attractivité du droit français. Les auditions ont toutefois montré que cette ordonnance était entaché d'un certain nombre d'imperfections incontestable et manifeste que notre rapporteur, a mis en évidence et dont la plupart lors de nos entretiens était reconnu et notamment par la chancellerie, le groupe lui ses partagent les propositions d'interprétation des dispositions du code civil issu de l'ordonnance, tout comme les amendements qui ont donc été adoptés en commission, ces propositions permettront véritablement de clarifier le sens de la loi paradoxalement aux commentaires parfois entendu qui craignent un pouvoir exorbitant d'interprétation du juge, j'ai été frappé par l'appel incessant des universitaires, mais également des magistrats de préciser à l'occasion de nous, de notre de nos débats, ces dispositions parfois floues, ces notions afin d'éclairer leurs interprétations et d'éviter d'éventuels préjudices aux entreprises l'approche retenue par notre collègue clarifie donc cette articulation entre droit commun et droit spécial, notamment en matière de clauses abusives ainsi l'article 1171 du code civil ne doit pas, selon nous, s'appliquer dans les champs déjà couverts par des articles du code du commerce ou du code de la consommation, elle précise les modalités d'application de la loi dans le temps, notamment dans les contrats renouvelés et les contrats prorogée. L'amendement modifiant l'article 9 complète certes précision en affirmant l'impératif de la de survie de la loi ancienne pour les contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance l'article 1195 du code civil est également amener amendé en privant le juge de son pouvoir nouveau pouvoir de révision du contrat, la commission des lois, met ainsi fin à une incertitude préjudiciable tant à la vie des organismes des entreprises qu'au droit français puisqu'il risque d'être écarté en raison de l'aléa économiques cette disposition porte en elle, ainsi les parties pourront toujours demander, d'un commun accord au juge d'adapter le contrat à défaut d'accord, ce dernier pourra y mettre fin, un mot sur la modification de l'article 1343 3 qui limite le paiement devise internationale au seul cas prévus par des contrats internationaux ou des jugements étrangers la modification opérée par nos collègues de la commission des lois, répond aux interrogations des acteurs économiques mais sur ce point, j'interviendrai au cours des débats pour évoquer le risque que représente aujourd'hui des facteurs comme l'extraterritorialité du droit américain, vous le comprenez, mes chers collègues, l'objectif de sécurité juridique pour nos entreprises, a nécessité de trouver un subtil équilibre entre stabilité d'un texte déjà en vigueur est nécessaire clarification attendue par les professionnels du droit.

Inès, comme l'ont dit un certain nombre de beaucoup de mes collègues pas acceptable que le Parlement soit ainsi sa saisie d'un projet de loi de ratification, un an après l'entrée en vigueur de l'ordonnance et on le voit bien aujourd'hui, ceci dans l'intérêt des entreprises et des acteurs du du droit, ce débat aurait dû se tenir en amont avant son entrée en vigueur, nous comptons donc sur votre gouvernement madame la ministre, pour impulser à l'avenir une stratégie plus constructive et respectueuse des missions confiées à chacun par les Français, contourner le Parlement, on le voit dans ce cas précis, c'est créer une situation d'insécurité donc de fragilité juridique dans sa sagesse, le disait : le Sénat fait aujourd'hui une proposition de loi de ratification qui va dans le sens à la fois des intérêts des entreprises et du droit français, mais nous espérons que cette méthode de passage en force ne se renouvellera pas et que nous pourrons, notamment à l'avenir sur le dossier du régime de la responsabilité contractuelle engager ensemble un travail législatif sérieux et partagé en amont. Le groupe UC demeure attentif aux réalités et aux besoins des acteurs économiques de notre pays et notamment aux petites et moyennes entreprises, vous l'avez dit Madame et ce qui est moins adapté face au bouleversement juridique occasionnés par cette réforme du droit des contrats, il sera vigilant au retour terrain aux effets collatéraux voire législatif que cette réforme pour révéler dans les prochains mois il suivra je l'dit notamment les effets internationaux au regard des objectifs affichés d'attractivité et de compétitivité du droit français mais aussi de perméabilité face à ce phénomène que j'ai cité Dexter d'extraterritorialité du droit américain, je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole maintenant est à monsieur Jacques Bigot pour le groupe socialiste républicain pour 10 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président, la commission des lois au vice-président, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, finalement, le Sénat aujourd'hui se montre bon enfant à l'égard du gouvernement puisque, alors même qu'il n'était pas favorable au transfert au transfert de compétences en n'autorisant par la loi d'habilitation du 16 février 2015 le travail considérable qui a été fait par les juristes par les membres du cabinet de votre prédécesseur, ainsi que par les directions, notamment la direction des affaires civiles, que je salue ici. Ne Sénat auraient pu aujourd'hui dire nous voulons ratifier revenir travailler et mode. C'est plein dans sa dans sa grande sagesse, sous le regard de Portalis bien évidemment, le rapporteur n'a pas proposé la même chose, mais en même temps vous aurez noté Madame la Ministre que depuis il y a des choses qui ont changé,

et il a trouvé que l'habilitation en matière de droit du travail était de or du possible et même au sein de l'hémicycle, des gens ont évolué, donc ceci sans doute explique cela

le code civil ne bouge pas, mais il a considérablement bougé par des lois spécifiques : le texte du code civil de 1804 n'est plus celui qui régit le droit du travail alors qu'il ne réagissait à la fin du 19ème siècle, dans les conditions que l'on connaît le texte du code civil ne réagit plus les beaux le de l'autre de la location d'habitations, les baux commerciaux, tout ça, il a bien fallu à un moment donné que le législateur intervienne pour protéger et le travail qui vient d'être fait qui nous est proposé aujourd'hui à la ratification et je pense qu'effectivement, il ne faut pas qu'on bouleverse trop les choses parce que de toute façon, les commentateurs juridique qui ont déjà fait leur cette ordonnance et qu'il comprendrait mal qu'on Vienne beaucoup la modifier, je pense même qu'il serait capable de critiquer l'attitude de Corée, le Sénat, monsieur le rapporteur, mais il n'empêche que le travail qui a été fait, mérite d'être salué, parce qu'il est le fruit de 10 années de réflexion, des techniciens, des spécialistes, des juristes, mais aussi des professionnels concernés, chambre de commerce, le MEDEF et d'autres qui ont été interrogées, et finalement il est aussi le fruit de la compilation et de la mise en oeuvre de ce que la jurisprudence a construit depuis de nombreuses années, cette compilation rendait nécessaire à un moment donné une clarification, elle était attendue, et le gouvernement qui a précédé celui auquel vous appartenez aujourd'hui a eu effectivement le courage de se lancer dans cette activité et d'enfin aboutir, on peut lui reprocher de ne pas être venu devant le Sénat avant mais finalement c'était pour laisser l'occasion d'en parler, madame la Ministre, cette évolution consiste aussi en l'abandon d'un certain nombres de de 2 concepts. Objectivement, pour les civilistes, la distinction subtile entre l'objet et la cause du contrat était devenue à peu près impraticable et difficilement explicable lorsqu'on faisait des cours de droit à à nos étudiants, donc on a bien fait de l'abandonner certains ont de la nostalgie, mais globalement, je pense que c'est pas utile, par contre, les principes qui sont affirmées ici reste nécessaire et fondamentaux : d'abord la notion de liberté contractuelle, ce qu'on appelait jadis l'autonomie la volonté doit rester dans le domaine des contrats l'action principale, le 2ème sujet que le monde économique, attend, c'est la sécurité contractuels, faire en sorte que l'on soit sûr que ce qui était écrit : rester sur un

parce qu'effectivement la loyauté contractuelle doit être un principe et et re-rappelé ce principe de la bonne foi, le décliner dans différents textes sur l'exécution du contrat et parvenir effectivement à ce que les juges lorsqu'ils seront amenés à trancher des contentieux vérifie à ce que la bonne foi soit respectée par les parties est important, il peut paraître regrettable que l'on n'est pas plus travailler au sein des du parlement sur ces textes parce que nous parlons beaucoup ici des enjeux économiques, or le droit des obligations, le droit des contrats et fondamental dans le monde économique et qu'a besoin de monde économique c'est de cette sécurité, je parlais à l'instant, c'est de l'efficacité des contrats. Et de ce point de vue là d'éviter des contentieux et des interprétations complexe mais c'est aussi la question de l'équité et sur la question de l'équité, nous aurons, nous aurions plusieurs sujets abordés, l'équité ne concerne pas que le faible à l'égard du fort Portalis en parler déjà l'équité, elle suppose aussi. Que l'on voit comment est construit un contrat enfin apparaît dans le texte du code civil maintenant la notion de contrat d'adhésion, notion qui a été construite par la jurisprudence, mais avec une énorme frilosité et on reste d'ailleurs encore sur ces sujets très philosophe parce que il suffit de regarder les résolutions du Conseil de l'Europe de 1976 sur les clauses abusives pour se rendre compte que il y a encore du chemin à parcourir, et que même les directives européennes ne nous ont pas aidés, a suffisamment construire à la lutte contre les clauses abusives mais forte heureusement dans le code civil désormais et cela va concerner aussi les petites entreprises qui sont souvent soumises à des contrats d'adhésion dans le monde économique dans un contrat d'adhésion toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et réputée non écrite, cela créé pour celui qui rédige le contrat d'adhésion, une incertitude sur la fiabilité de son contrat, et s'il veut que son contrat soit sur il a intérêt effectivement à ce qu'il soit équilibré. Dans ce même domaine. L'ordonnance ouvre et on va en parler à propos des amendements un Champ nouveau sur la question de l'imprévisibilité d'un événement qui fait que l'exécution du contrat. Pour émettre une des parties en défi voire même rendre l'exécution du contrat difficile. Quelle doit-être à ce moment-là le rôle du juge est-ce que le juge doit simplement, comme le propose autre rapporteur constater qu'il n'y a pas d'accord entre les parties et à la limite, tenu qu'on ne compte tenu de la situation, prononcé la résiliation, la résolution du contrat on peut-il aller jusqu'à la révision, il faut sans doute permettre d'aller jusqu'à la révision parce que l'intérêt des parties et l'intérêt et leur intérêt économique et de réussir mais qu'est-ce qui va pas se passer, monsieur le rapporteur, sinon match. Non, ce qu'ont prévu les auteurs de la ambiance, va pouvoir jouer un rôle de conciliation écoutez les parties construire à partir de cette saisine donc permettre à l'une des parties de saisir le juge. Pour une demander de modifier et de réviser le contrat me paraît aussi utile que de simplement lui permettent de le résilier parce qu'il n'est pas forcément de l'intérêt des parties de le résilier, donc vous aurez compris, madame la ministre, que notre groupe va, comme je pense la majorité des sénateurs aujourd'hui tout en ayant, regrette l'habilitation à Benicio suivre le travail qui a été fait dans vos services approuvés pour Lens pour l'essentiel vautrant romance fait faire en sorte du coup qu'il n'y a pas d'insécurité juridique pour les partenaires au contrat qui ont signé des contrats soumis à à cette ordonnance depuis le 1er octobre 2016 et puis en même temps savoir que rien n'est terminé, que les parlementaires ont fait leur travail. Sous contrainte, mais que la jurisprudence continuera à faire en sorte que le droit évolue parce que bien évidemment les textes ouvrent toujours plein interprétation et nous le verrons bien à l'avenir, donc les commentateurs ont encore du travail peut-être nous aussi. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Alain Marc, pour le groupe RTL il pour 6 minutes. Madame Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mais, chers collègues, je vais en préambule, reprendre une citation archi-connu ma vraie gloire n'est pas d'avoir gagné 40 batailles à Waterloo effaceras le souvenir de tant de victoires, ce que rien effaceras ce qui vivra éternellement, c'est mon code civil. Formule 1 c'est vous d'éternité Napoléon ne croyait pas si bien dire puisque plus de 200 ans après l'héritage de son code civil est toujours là. L'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations a toutefois procéder à une refonte d'ampleur du code civil en consolidant modernisant et clarifiant endroit défraîchis, sans pour autant le bouleverser ni constituer une rupture en 2015 le Sénat tout entier s'était opposés à ce que le gouvernement procédera par ordonnances à la réforme la plus ambitieuse du code civil depuis 1880. Il y a un an, le 1er octobre 2016, l'ordonnance est entrée en vigueur lors des travaux en commission, il est apparu particulièrement l'important de ne pas créer un droit intermédiaires qui ne s'appliquerait qu'aux contrats passés entre octobre 2016 et la promulgation de la loi de ratification afin d'éviter de faire un coup exister 3 régimes mesures juridiques simultanément, c'est pourquoi le rapporteur François Pillet a estimé qu'il fallait ratifier l'ordonnance sa modification majeure. à l'avenir, d'ailleurs, il serait souhaitable que les ordonnances soient soumises à ratification avant leur entrée en vigueur il y va élire et de la stabilité du droit. Cette réforme de grande ampleur du droit des contrats et des obligations effectué par ordonnance sera suivie d'une toute toute aussi grande réforme du droit de la responsabilité civile qui fera quant à elle l'objet d'un projet de loi, ce dont on peut tous se féliciter, globalement, cette réforme du code civil, M. pacte le droit des contrats sur 2 points : d'une part et le codifie les acquis de la jurisprudence, d'autre part, et le réorganiser les dispositions du code à l'intégrer certaines innovations et un supprimant certaines notions. Les consécrations changements ainsi opérée par la réforme du droit des contrats sont particulièrement important parmi ceux-ci, on peut relever la disparition formelle de la clause de l'accord, la sanction des clauses abusives dans les contrats d'adhésion, la violence, par abus d'un état de dépendance les demandes faites sous forme interrogatoire le maintien du contrat comme sanction de sa mauvaise information, l'intégration de la théorie de l'imprévision l'exception pour une exécution à venir la paralysie de l'exécution forcée en cas de disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier la faculté de remplacement sans autorisation du juge ou encore la modification de la hiérarchie des différents mécanismes de résolution pour inexécution après avoir examiné le rapport de François Pillet sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance du 10 février 2016, la commission des lois adoptées 14 demande de clarification de précision ou de mise en cohérence essentiellement. Ainsi, la Commission a précisé la définition du contrat d'adhésion et le charme de la secte de la sanction des clauses abusives dans ses contrant ainsi que les critères autorisant le paiement en devises sur le territoire français. L à mieux articuler les règles en matière de capacité et de représentations avec le droit des sociétés, elle a supprimé le pouvoir de révision du contrat par le juge en cas de changement même imprévisible de circonstance, enfin, elle a affirmé clairement que cette loi nouvelle ne doit pas s'appliquer aux contrats conclus antérieurement par ailleurs, la commission des lois, apporter un certain nombre de clarifications concernant notamment la distinction entre règles impératives et supplétive et l'articulation entre droit commun et droit spécial avant de conclure : je souhaite remercier à cette tribune, le rapporteur de ce texte, notre collègue François Pinault le travail qu'il accomplit sur une texte aussi volumineux est colossal cette réforme du Kossi ville apparaissant nécessaires et la commission ayant apporté au texte les corrections de nature à répondre aux critiques les plus fondés et légitimes, le groupe République et Territoires et les indépendants votera en faveur de la ratification de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations. Lègue la parole maintenant état Madame Maryse Carrère pour leur groupe RDSE.

Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, lors de la publication de l'ordonnance du 10 février 2016, beaucoup ont rappelé le défi particulier de porter des modifications au Code civil un texte en raison de la fierté comme tiré Napoléon l'imminence de ces prestigieuses auteur et le poids des années écoulées pendant des siècles, en effet, le syndrome de la main tremblante par Montesquieu a tenu le livre 3 du code hors de portée du législateur, il s'agit donc de féliciter ceux qui, à la suite du professeur Cathala se sont attelés à cette tâche fastidieuse et exigeante. Une actualisation était nécessaire l'évolution parallèle des droits de la consommation, de la concurrence d'une part et de la jurisprudence en matière civile, d'autre part, ont généré un autre défaut dénoncé par l'auteur des Lettres persanes que je cite quelques heurts ont affecté de se servir d'une autre langue que la vulgaire absurde pour un faiseur de lois, comment peut-on les observer si elles ne sont pas connus, de même le maintien des règles éparses contestables, comme le sont les constructions jurisprudentielles faisait obstacle à une application sereine du droit. Cependant, si nous nous contentions de ratifier des ordonnances au seul motif qu'elle codifie à droit constant, sans analyser les règles dégagés par la jurisprudence ainsi érigée en loi ni se laisser la possibilité d'un débattre nous manquerions notre devoir de législateur lors de notre examen du texte au sein du groupe RDSE, nous avons veillé à ce que les modifications introduites ne Sédunois n'y a pas de l'esprit de 1804 telle que résumée par Portalis lors de son discours préliminaire du 1er projet de code civil : un homme qui traite avec un autre homme doit être attentifs et sages, il doit veiller à son intérêt, prendre les informations convenable et ne pas négliger ce qui est utile, l'Office de la loi et de nous protéger contre la fraude d'autrui, mais non pas de nous dispenser de faire usage de notre propre raison, c'est pourquoi nous voyons d'un bon oeil toute évolution tendant à situer l'individu contractant dans le Champ de la rationalité plutôt que de la moralité par essence évolutive, la promotion du principe de la liberté contractuelle et la suppression de bonnes moeurs comme limite à ce principe sont des évolutions essentiel la liberté contractuelle en ressort renforcé seule s'impose à elle, le respect de l'ordre public et des droits et libertés fondamentaux réputé immuable : l'effort d'actualisation est incontestable, il se manifeste par la suppression des anachronismes tels que la notion de bonnes moeurs que j'évoquais à l'instant, ou encore de celle de gestion en bon père de famille, pour l'heure, leur utilité juridique n'étant plus évidente de la même façon sont insérés dans les livres 3 de nouveaux concepts, adapté à la transformation de la pratique contractuelle, tels que les contrats d'adhésion ou les camps contrats conclus par voie électronique, il couvre aujourd'hui une part substantielle des échanges économiques sur notre territoire, le rescrit Psion 5 du code permet plusieurs clarification qui nous semble aller dans le bon sens. a un est ainsi aussi de la protection contre les clauses abusives d'un contrat d'adhésion qui ne s'applique plus seulement aux consommateurs, mais à tous les souscripteurs de ce type de contrat, il en est ainsi également des dispositions qui font rentrer des règles relatives au contrat électronique dans le droit commun, plus de 15 ans après la directive européenne sur le commerce électronique. Il faut à ce propos, saluer le renforcement de la protection de la partie faible qui a entériné, parfois même en dépasse les équilibres jurisprudentielle existants, nous considérons ainsi que l'introduction de la théorie de l'imprévision du code civil, permettra d'apaiser les relations contractuelles en garantissant mieux l'équilibre financier du contrat, la création d'un devoir général d'information procède de la même logique conforme à les prix à l'esprit de 10804 que j'évoquais à l'instant, protégé, c'est sanctionner la fraude mais également la prévenir, bien entendu on ne réécrit pas près de 300 articles Saint-Cricq quelques incertitudes et certains jeux ajustements seront peut-être nécessaires par la suite, en fonction de la portée : donner à telle ou telle disposition, je pense notamment à la définition de la dépendance économique dans l'ensemble, nous sommes donc très favorable à la ratification de cette ordonnance qui modernise notre droit de contrat, des contrats et des obligations, tout un intégra en code civil une partie de l'acquis des droits des consommateurs. à l'approche des débats budgétaires nous inquiétudes sont ailleurs, comme ses prédécesseurs ce gouvernement semble faire le pari que le renforcement de la sécurité juridique permettra à lui seul de réduire les recours au juge et de désengorger les tribunaux, la situation budgétaire de l'autorité judiciaire est pourtant devenue si critique qu'elle surgit en toute occasion et qu'elle est désormais présenté comme un obstacle à la mise en place de chaque réforme, nous considérons qu'à l'avenir des moyens supplémentaires devraient être réservés pour accompagner l'adaptation des magistrats à de telles évolutions législatives dans un souci de bonne administration de la justice, une fois exprimé cette réserve les membres du groupe RDSE voteront en faveur de la ratification de cette ordonnance. Merci, cher collègue. La parole maintenant est monsieur Arnaud de Belenet pour la République en marche pour 6 minutes.

madame la garde des Sceaux, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, c'était évidemment avec l'humilité qu'induit la jeunesse de mon mandat, que je salue l'aboutissement du long processus processus de refonte du droit des contrats avec la proposition de ratification qui serait hautement responsable par notre assemblée de ce texte majeur est attendu ce texte marqué par la ténacité de la chancellerie et le travail considérable effectué ici singulièrement par notre rapporteur François Pillet et notre collègue Thani Mohamed soit affirme notre travail tradition civiliste et répond aux questions de sécurité juridique d'imprévisibilité d'accessibilité déficiences de cohérence européenne et d'équilibre des droits des contrats, mais aussi d'attractivité, je pense à l'attractivité du droit français, du point de vue strictement économique vis-à-vis des entreprises, mais aussi du point de vue de l'influence du système juridique français à l'étranger. Toutefois, compte tenu de la jeunesse de son application on tirer vanité à ce stade de parler sans mesure d'une meilleure attractivité de notre droit des contrats nonobstant cette incertitude: cette réforme est largement approuvée par les universitaires et les praticiens du droit, la nouvelle organisation des dispositions qui suivent l'avis du contrat répond à un souci de lisibilité nécessaire sa rédaction plus contemporaine améliore sans conteste sa compréhension la consécration de la liberté contractuelle de la force obligatoire du contrat du respect de l'ordre public et de la bonne foi garantissent un cadre cohérent et clair. Au-delà de la codification de la jurisprudence, le texte innove par plusieurs aspects, à commencer par la suppression de la cause du contrat, il adapte notre droit à la réalité de l'expansion du numérique, il apporte des précisions ou déconsidérés des consécration 11 utile pour les acteurs économiques comme le Champ de la capacité des personnes morales, l'acquisition de contrats ou de cessions de dettes pour les entreprises, par exemple. Le travail mené au Sénat. Confirme la formule de Guy Carcassonne, le tamis parlementaire a des vertus intrinsèques et sur le sujet particulièrement ardue et peu prospère politiquement est le droit des contrats, la commission des lois a ainsi adopté plusieurs modifications d'une grande technicité et précision de clarification substantielles, voire essentiel, avec notamment la clarification et la bilatérales isolation des définitions respectif du contrat de gré à gré du contrat d'adhésion, l'exclusion de la perte de chance des préjudice réparable. La détermination du fameux délai raisonnable susceptible à défaut d'interprétation, nous sommes attachés assez de moi la plus grande cohérence du régime de la réticence de l'et de celui de l'obligation d'information pré-contractuelle et bien sûr la saisine du juge en cas de prix abusifs, non seulement pour obtenir des dommages et intérêts venant indirectement réduire le montant du prix mais aussi la résolution du contrat pour couvrir l'hypothèse où l'exécution de celui-ci n'est pas achevée mais aussi la réduction de l'aléa judiciaire introduit par l'ordonnance sur le contentieux de la réduction de du prix par exemple. Permettez-moi 2 2 dernières illustrations de ce travail mené ici l'autorisation du paiement en monnaie étrangère, d'une obligation de sommes d'argent payé en France et le règlement de la question essentielle de l'application dans le temps de la loi, je note enfin l'affirmation par notre rapporteur d'un certain nombre de 2 points qui permettront au juge. De ne pas laisser prospérer une jurisprudence nombreuses controversé et multiple sur un certain nombre de points en commission et ici même, comme vous l'avez fait tout à l'heure, notamment sur l'information elle sur la confidentialité de l'information et sa définition au regard de l'intégration des travaux de notre assemblée, nous appellerons à la ratification, responsable de cette réforme. Merci, cher collègue, la parole est désormais à Madame Muriel Jourda pour les républicains pour sa minute.

Madame la présidente, madame la garde des Sceaux du rapporteur, mes chers collègues, comme cela vous a été répétée à l'envi depuis tout à l'heure, nous sommes réunis ici pour débattre d'un projet de réformes ambitieux de notre droit civil un projet nécessaire qui est l'aboutissement d'une longue réflexion relative à l'adaptation de notre endroit où notre droit aux enjeux économiques contemporains. Comme vous le savez, le droit des obligations que nous connaissons aujourd'hui est issu de la lettre du code civil, mais aussi d'une jurisprudence abondante qui a fait grandement évoluer notre droit depuis 1804 le droit des obligations repose en partie sur un vaste corpus de jurisprudence, alors même que notre droit est issu d'une tradition civiliste aux règles écrites et codifiées cette particularité est source de grands travaux intellectuels et doctrinaux mais rend délicate aussi la lisibilité et la prévisibilité de notre droit, pourtant essentielle aux acteurs économiques, la réforme était donc nécessaire, pour ce faire, la chancellerie a publié en février 2015, un avant-projet d'ordonnance portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations soumis à contribution publique ce projet a suscité de très importantes contributions et prend sa source dans les nombreux travaux de la doctrine en France et des projets d'harmonisation européenne du droit des contrats l'objectif 1er de ce projet de réforme telle que présentée dans le rapport au président de la République et de renforcer la sécurité juridique du droit des contrats. Comme l'indiquait notre rapporteur, cet objectif est primordial, il est en grande partie atteint en effet la nouvelle rédaction qui a vocation à intégrer le code civil et plus clair et l'organisation du code plus didactique, renforçant grandement sa lisibilité ainsi un nouveau chapitre introductif rappelle clairement les principes directeurs du droit des contrats par ailleurs la réforme renforce la cohérence de notre droit des contrats en codifié dans la jurisprudence de la Cour de cassation, les auteurs de cette réforme ont permis en réalité à l'intégralité du droit positif de rejoindre le code civil, la réforme marque aussi une évolution majeure introduisant dans le code civil des innovations juridiques à la portée nous négligeables je pense bien sûr à la théorie de l'imprévision, soit de la police, possibilité pour le juge d'intervenir dans un contrat en cours dans certaines conditions, nous y reviendrons tout à l'heure, je pense, je pense aussi à la violence économique nouveau vice du consentement ou encore aux nouvelles actions dites interrogatoire comme en matière de pacte de préférence ou d'action en nullité qui permettent une meilleure information des partis. La commission des lois du Sénat a choisi la ratification de cette ordonnance, qui a fait l'objet d'un bon accueil de la part de la doctrine également des praticiens. praticiens. En dépit de la qualité générale de sa rédaction. Nous devons rappeler que ce processus de réforme du droit des obligations telles qu'il s'achève aujourd'hui. Et marquée par un certain mépris du rôle du législateur, je n'oserais pas dire un mépris certain. En effet, il faut rappeler l'opposition ferme du Sénat à la méthode des ordonnances en particulier s'agissant de cette réforme. Lors de l'examen de l'habilitation demandée par le gouvernement. Le Sénat avait souligné l'importance d'un débat public sur une réforme de cette ampleur. Le choix de recourir à la méthode des ordonnances avaient de fait grandement limiter les possibilités de débat au sujet d'une réforme aux innombrables conséquences pour la vie économique du pays. On rappellera que telle réforme ne se borne pas importer des questions d'une grande technicité. Le droit des obligations soulève des interrogations d'ordre politique. Telle que la tension entre un impératif de justice dans le contrat et le respect de l'autonomie des partis, et plus généralement de la sécurité juridique des conventions. Enfin que dire du manque de cohérence, s'agissant de la volonté du gouvernement de d'y joindre la réforme du droit des contrats de celle du droit de la responsabilité civile pourtant inextricablement liés, le choix de recourir à cette méthode dessert, de toute évidence, les objectifs de la réforme, la marge de manoeuvre du Sénat pour modifier les dispositions issues ordonnance est plus que limitée, comment remettre en cause les fondements d'un texte auquel les praticiens se sont préparés et désormais adapter cette assemblée ne peut transformer les dispositions issues d'ordonnance endroit transitoire, sauf à créer encore plus d'insécurité juridique au détriment des objectifs de sa très. Pour autant, la commission des lois a choisi de ratifier l'ordonnance tout en apportant de nécessaire et justement de clarification de textes ces correctifs permettent notamment d'évacuer plusieurs ambiguïtés importante et de préciser les modalités d'application de la nouvelle loi aux contrats en cours pour l'ensemble de ces raisons, tout en déplorant la méthode choisie par le gouvernement, le groupe Les Républicains votera en faveur du texte de la Commission. Merci, cher collègue. La parole est maintenant Madame la Garde des Sceaux. Merci madame la présidente, simplement quelques quelques observations très rapides, en réponse à ce que les uns et les autres avaient évoqué l'un d'entre vous a dit que le Sénat était bon enfant. Je ne reprendrai pas cette expression-là que je trouve un peu, comment dirais-je, familière, j'ai plus de respect pour le Sénat, que de le considérer simplement comme bon enfant, je crois au contraire que le Sénat fait preuve ici de. en nous, en ayant habilité le gouvernement a travaillé sur ce sujet et j'ai dit à quel point la concertation qui avait été conduite le travail qui avait été menée avec de très nombreux experts a permis d'aboutir au texte qui vous est aujourd'hui soumis, et donc cette une manière de montrer que le travail qui a été accompli est extrêmement sérieux et de votre part soumettre ce texte à ratification constitue également une marque de respect pour le Sénat, bien entendu, qui est tout à fait naturel, je dois dire, face aux critiques que beaucoup d'entre vous ont formulé sur la technique des ordonnances et de l'article 38 c'est une technique qui est constitutionnel est expressément prévu par notre texte fondateur et à partir du moment où le fait le choix de revenir de manière explicite devant vous, par un texte autonome, il me semble que c'est une manière d'écrire le texte de loi qui est tout à fait et performante et conforme à notre constitution et respectueuses de votre assemblée, et donc je crois que cette procédure là ne méritent pas l'opprobre dans laquelle vous la tenez sur le fond des points qui ont été abordés quelques expressions simplement Monsieur Collombat, merci infiniment pour votre soutien à ce texte et d'ailleurs, votre soutien également à plusieurs amendements ou le le gouvernement sera en phase avec vous, pardon, sur un certain nombre, oui, oui, je tiens à le dire sur plusieurs amendements, j'ai bien noté, bien que j'ai trouvé que ce soit un petit peu éloigné, mais enfin, j'ai pris bonne note de vos observations qui ont d'ailleurs été également formulée par l'une d'entre vous, sur le budget de la justice, c'est peut-être un peu loin du sujet qui nous occupe, mais je comprend vos préoccupations, j'aurai l'occasion de revenir devant vous pour vous exposez que le budget de la justice en 2018 augmentera de 4 pourcent de de presque 4 pourcent il il en sera de même sur les années 2019, 2020, donc j'espère ainsi que nous pourrons effectivement palier progressivement les difficultés que rencontre notre ministère et cela témoigne de l'effort que le gouvernement fait en faveur faveur de la justice à Madame Anne-Catherine loisirs et Fouzia vive raison de souligner qu'il y avait urgence à adopter cette réforme, et je vous remercie également pour votre soutien ainsi que celui de votre groupe, c'est effectivement un équilibre entre la modernité et le respect de nos principes constitutionnels, et il me semble que ce texte, je crois, peut jouer un rôle en faveur de l'attractivité de notre droit, j'ai été souvent extrêmement par par les rapports qui sont publiés sous l'intitulé doing Business chaque année et qui montre la place certes qui progresse, mais pas encore suffisamment de la France parmi l'ensemble des États dans le monde des affaires j'ai une certaine peut-être méfiance par rapport à ces rapports de la Banque mondiale, mais malgré tout, ils sont très significatif et je crois que si nous voulons être attractif, nous avions tout intérêt à revoir ce droit des contrats, c'est ce que nous avons fait, j'espère qu'avec d'autres mesures comme l'installation de la juridiction du brevet en France, comme la possibilité pour certaines de nos juridictions de traduire nos actes juridictionnels en anglais, je pense que tout cela contribuera puissamment à l'attractivité de la place de Paris et c'est tout à fait important je voudrais d'ailleurs toujours à Madame Loisy et soulignée parce que vous avez observé également le le délai l'importance du délai mis à demander la ratification de l'ordonnance devant vous, je voudrais dire ici que il faut bien entendu tenir tenir compte de la période électorale qui n'a pas permis de présenter ce texte devant vous auparavant et je vous ferai observer qu'il s'agit du 1er texte que le ministère de la Justice, présente lors de la 1ère session ordinaire ouverte depuis les élections de ce printemps. Monsieur Bigot, vous êtes revenu sur la méthode et vous avez souligné le courage qu'il fallait pour s'attaquer à cette immense question du droit des contrats et des obligations, il en fallait, en effet, je revois remercie d'ailleurs pour ce que vous avez dit et notamment sur la question de l'imprévision et du rôle du juge je crois. Que c'était une novation tout à fait importante qui a été ainsi traduite mais vous avez eu raison également de dire que l'histoire ne s'arrête pas là et que la question notamment qui viendra de l'interprétation de certaines de nos dispositions par le juge de la manière dont les entreprises et les acteurs vont s'emparer de ce texte construira cette histoire et fera vivre cette nouvelle étape de notre code civil, monsieur le sénateur Marc, je vous remercie également de vos observations et je salue votre sens de la mesure et votre soutien au texte, ainsi que celui. Du groupe que vous représentez, enfin, à Madame Carrère, j'ai apprécié vos propos sur le souci que la rationalité l'emportait dépasse les émotions et c'est vrai que ce traité ce texte traduit bien cela, effectivement, vous avez également évoqué la question question du budget de la justice, je ne reprends pas ce que j'ai dit aux sénateurs Colomba vous avez souligné l'intérêt d'accompagner cette réforme également, je dois dire, de ce point de vue qu'il y a plusieurs éléments qui permettent l'accompagnement de cette réforme, j'ai souligné dans mon propos introductif, le rapport du président de la République, le le rapport au président de la République est extrêmement épais et qui est à une forme de de vade-mecum des fiches techniques également qui ont été élaborés qui seront mis à disposition des magistrats, des formations qui seront faites au sein de l'École nationale de la magistrature, qui ont déjà commencé d'ailleurs et également diverses présentations de la réforme aux juridictions. à monsieur Debré, le nez, j'ai été particulièrement sensible à l'hommage que vous avez rendu à mon collègue Guy Carcassonne j'ai j'ai été très touchée de ce que vous avez dit, et je vous remercie également du soutien du groupe, la République en marche enfin Madame Jourdain je crois que vous avez eu raison Madame la sénatrice de souligner que c'est une réforme qui, globalement, avait été a été très bien accueilli par la doctrine, même si des inflexions, des commentaires ont été apportées, ce qui est tout à fait naturel et nous allons d'ailleurs dans une certaine mesure, tenter de répondre à quelques-unes des observations qui ont été formulées, je vous ai répondu tout à l'heure sur le terme mépris que vous avez utilisé, je ne pense pas qu'il y ait aucun mépris du gouvernement à l'égard du Parlement, c'est pas que je ne pense pas d'ailleurs ce que j'en suis certaine et le fait que je sois aujourd'hui devant vous, pour travailler avec vous sur ce texte me semble être exactement le contraire du mépris, mais le souci bien sûr de respecter vos compétences, voilà ce que je vous les évoquez nous aurons effectivement à retravailler ensemble autour de la responsabilité, car c'est le dernier chantier du code civil qui nous reste à revoir et nous aurons l'occasion de repenser avec vous et les modalités et le contenu de ce texte, je vous remercie. Merci Madame Lagarde sous la discussion générale est Close, nous passons la discussion du texte de la Commission,

Merci madame la présidente, il s'agissait simplement de préciser la notion de de contrats exécution successives pour prendre en compte un certain nombre de de prestations qui par nature ne qui par nature ne peuvent s'exécuter que dans la durée. Comment, contrat de travail ou location d'un bien, mais c'est un amendement a fait l'objet d'un retrait

afin de restaurer l'attractivité du droit français des contrats et le rendre plus efficient pour nos entreprises, en particulier nos PME, je proposerai 9 amendements et c'est le 1er d'entre eux. Le nouvel article 1112 tirer 1 du Code civil introduit un devoir général d'informations d'ordre public, ce devoir d'information est subordonné à plusieurs conditions, l'importance déterminante de l'information pour le consentement de l'autre partie, la connaissance de l'information par le créancier l'ignorance de l'information par l'autre partie cette ignorance devant être légitimés pouvant tenir aux relations de confiance entre les co-contractants le droit comparé nous apprend que de nombreux autres systèmes juridiques impose une obligation de se renseigner. Toutefois, le devoir de se renseigner, ne saurait annihiler totalement l'obligation d'information, il reviendra aux juges de trouver un juste équilibre entre ces 2 obligations aussi le devoir de se renseigner visés par le présent amendement n'a pas pour objet de supprimer l'obligation d'information mais d'inciter le juge à tenir compte de la situation particulière des partis. Oui, madame la présidente, lors des auditions que comme j'ai mené cette question du devoir de s'informer comme corollaire de la nouvelle obligation d'information pré-contractuelle a bien été soulevée en effet que jamais tenu compte dans le rapport, je reviens sur ce point parce que c'est le 1er amendement que nous discutons pour rappeler l'attention du Sénat sur un point, à l'occasion de cette discussion, à l'occasion de la ratification de cette ordonnance est proposé à la Commission de modifier l'ordonnance lorsque c'était indispensable et sinon de délivrer une interprétation claire et incontestable, et la semaine dernière, la Commission a validé ses interprétations au titre des travaux préparatoires qui encore une fois, sont source de droit et et ce qui va éviter beaucoup de modifications du taff de l'ordonnance qui ne portait que sur des questions d'interprétation sur lesquels d'ailleurs, nous étions quasiment tous d'accord, cet amendement entrent dans dans ce cas, ainsi pour faire naître l'obligation d'information, celle-ci doit être, c'est dans le texte, déterminante pour le consentement de l'autre partie, mais cette dernière doit aussi on ignorait légitimement l'existence ou faire confiance à son compte il faut déduire du critère de l'ignorance légitime de l'information par le co-contractants que le texte consacre bien un devoir de s'informer, ce que confirme d'ailleurs le rapport au président de la République qui indique bien que le devoir de sa forme et fixe la limite de l'obligation précontractuel de l'information ainsi d'un côté, lorsque l'information était cibles pour le con contractant seniors en ce ne sera plus légitime et de l'autre côté, lorsqu'un lien de confiance particulier existe, voire très existe entre les 2 parties, cette situation peut à l'inverse, justifier une obligation d'information particulière, l'objet de l'amendement m'apparaît donc satisfaits par l'article telle qu'il est rédigé et au regard de l'interprétation que je vous propose expressément de lui donner donc si vous le souhaitez, cet amendement, sinon un avis défavorable. L'avis du gouvernement, Madame Lagarde sont. Oui, madame la présidente, je partage l'avis de monsieur le rapporteur, l'une des innovations de l'ordonnance a été l'introduction dans le code civil d'un devoir général pré contractuelle d'information qui étaient déjà consacré pour une large part par la jurisprudence, madame la sénatrice, je tiens à vous rassurer ce devoir d'information trouve bien sa limite dans le devoir de s'informer de l'autre partie s'il n'est pas expressément inscrit dans le texte, il s'en déduit toutefois la définition du devoir d'information telle qu'elle résulte de l'ordonnance prend déjà en considération une obligation pour l'autre partie de se renseigner en effet le manquement au devoir d'information ne peut être sanctionnée que si l'ignorance de celui qui s'en prévaut et légitime à cet égard, ne sera donc légitime à ignorer une information essentielle que celui qui serait dans l'incapacité d'y accéder, seul l'ordonnance n'a pas pour objet de déresponsabiliser les co-contractants, tout au contraire, les relations qui unissent une partie à son co-contractant peuvent également dans certaines circonstances, justifier qui lui fasse une confiance particulière, par exemple, si je suis associé dans la société, dont l'autre partie et dirigeant social je peux légitimement penser qu'il m'a communiqué les informations sur la situation financière de la société, de se renseigner, sera ainsi moduler selon la nature de l'information et selon la qualité respective des partis, c'est la raison pour laquelle, à l'image de ce qu'a fait monsieur le rapporteur, je vous propose soit de retirer l'amendement sinon chance solliciterai je serais défavorable. Madame Mellow voulez. Merci madame la présidente, je vous remercie, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur pour les précisions que vous venez d'apporter et je retire l'amendement. nous allons donc passé toujours après l'article 3 à un amendement additionnels qui est le média moment numéro 27 présenté par Monsieur de Belenet.

monsieur Vernet, nous allons passer à l'article IV je suis saisi d'un amendement numéro 13 présenté par le gouvernement. Madame Lagarde est souvent présenté cet amendement. Oui, madame la présidente, l'article 1117 prévoit que l'offre de contracter. Devient caduc en cas d'incapacité ou de décès de son auteur, avant son acceptation la commission des lois a souhaité étendre cette solution en cas de décès du destinataire de l'offre, cela ne me semble pas opportun le lien inextricable entre l'offre de contracter et son auteur justifie effectivement qu'elle n'engage pas ses héritiers, en revanche, rien ne justifie qu'une offre de contracter prennent systématiquement, enfin, au décès de son destinataire, la jurisprudence a pu sembler en ce sens, aller en ce sens, mais une telle solution a été critiqué, à juste titre par la doctrine une telle caducité Deloffre peut se comprendre lorsque le contrat projeté est un contrat, une suite eu personne et c'est-à-dire que la personne du co-contractants est déterminante, je vous donne un exemple : si j'ai adressé une offre de prestations à un professionnel pour la qualité de son travail, il est logique que son décès rende mon offre caduque, en revanche, dans d'autres types de contrats, la personne du co-contractants n'est absolument pas déterminante et l'offre de contrat doit pouvoir être transmise aux héritiers ainsi l'offre de vente qui est faite au propriétaire de l'appartement mitoyen pourrait être acceptée par son héritier s'il décède avant d'avoir accepté, c'est pourquoi je vous invite à revenir au texte initial pour laisser la jurisprudence apprécier la solution la plus opportune, selon le type de contrat proposé. proposé. Le rapporteur pour la commission. Madame la présidente de la commission des lois, qui a revu tous ses amendements, ce matin, donné un avis défavorable je m'explique sur les raisons de celui-ci, le texte de la Commission prévoit la caducité de l'offre en cas décès du destinataire, eu égard à une jurisprudence, vous venez de la citer selon laquelle qui est constante selon laquelle l'offre ne se transmet pas aux héritiers, certes, comme vous l'avez dit exactement certains auteurs avancent que l'offre ne deviendrait effectivement caduque, que si le contrat a projeté était intuitu persone et, ce qui signifie qu'il était fait en considération d'une personne, toutefois, la doctrine est d'ailleurs pas tout à fait unanime sur ce point, mais surtout le silence de la loi constitue une source d'incertitude juridique pour les héritiers se trouvant dans cette situation, qui vont être obligés de s'en remettre aux tribunaux après le décès d'un proche, ce qui ne me semble pas satisfaisant, vous l'évoquez d'ailleurs le recours aux tribunaux dans la motivation de votre amendement, mais ce sont précisément les raisons pour lesquelles la commission a souhaité clarifier explicitement ce point dans l'article 1117 du code civil, afin de garantir un régime de Loft protecteur et stable pour les partis, c'est-à-dire en fait de donner une sécurité juridique par un texte très précis, c'est la raison très technique de cet avis défavorable. Nous avons donc passé aux explications de vote Monsieur Bigot. Bigot. Le ministre nous suivrons l'avis du rapporteur parce que on a dit tout à l'heure qu'on a besoin de sécurité juridique, il est important pour l'auteur de l'offre d'avoir une sécurité son contractant

Ce qu'il y a d'autres explications de vote, donc je vous rappelle l'avis défavorable du de la commission évidemment l'avis favorable du gouvernement et je vais donc soumettre au vote de l'amendement numéro 13 qui est pour. Qui est contre. L'amendement n'est pas approuvé, nous allons donc passer un 2ème amendement du gouvernement que l'amendement numéro 14 madame la garde des Sceaux. Madame la présidente, il s'agit de l'article 1123 alinéa 3 du code civil. Cet article envisage l'hypothèse où un tiers qui s'apprête à conclure un contrat a un doute sur l'existence d'un pacte de préférence que l'autre partie aurait consenti et qui seraient donc susceptibles de violer en effet si l'autre partie avait déjà. Promis de proposer prioritairement le contrat à quelqu'un d'autre, la transaction risquerait d'être remise en cause. Le texte permet pour sécuriser donc la transaction dont il est question que ce tiers met en demeure le bénéficiaire présumé du pacte de confirmer ou non l'existence du pacte de préférence et d'indiquer s'il entend s'en prévaloir, s'il répond négativement ou, à défaut de réponse dans le délai accordé par le tiers le bénéficiaire ne pourra plus ensuite agir en nullité du contrat, ce dispositif est donc porteur de sécurité juridique. Le tiers doit fixer un délai de réponse dans sa mise en demeure qui doit être raisonnables imposé dans la loi, comme le souhaite donc la commission que ce délai soit de 2 mois ne permettent pas selon le gouvernement, d'adapter la durée du délai aux circonstances, or selon la complexité du contrat projeté le bénéficiaire peut avoir besoin de temps plus ou moins le plus ou moins long pour évaluer s'il a intérêt à se prévaloir du pacte que l'on songe par exemple. Le franchiseur avec lequel le franchisé s'était engagé à contracter en priorité s'il vendait son entreprise s'il est interpellé par un tiers, auxquels le franchisé a proposé son entreprise le franchiseur doit pouvoir examiner l'opportunité du rachat sur un plan juridique financier opérationnel et les conditions mêmes de ce rachat, un délai de 2 mois pour être alors paraître inadaptée car insuffisamment long à l'inverse, dans certaines situations, la transaction doit se faire rapidement et ne nécessite pas, ne présente pas difficulté le délai de mois pourra être trop long, je vous invite donc à bien vouloir revenir au texte initial qui je vous le rappelle, exige simplement que le tiers fixe un délai de réponse aux bénéficiaires présumés du pacte l'exigence du caractère raisonnable de cette, de ce délai permet en cas de contentieux que le juge s'assure que le délai fixé était bien n'adapté aux circonstances. Monsieur le rapporteur pour la commission. Président de la com mission des lois, c'est évidemment montré favorable à l'introduction des nouvelles procédures d'action interrogatoires qui vise à faciliter la vie du contrat Quid des délais raisonnables, certains délais raisonnables qui ont amené la Cour de cassation, dans un délai qu'il l'était beaucoup moins à rendre une jurisprudence constante au bout de 10 ans concernant l'action interrogatoire exercée par un type interroge la réaction interrogatoire exercée par un tiers dans le cadre du pacte de préférence qui fait donc l'objet du présent amendement, la commission des lois a souhaité préciser sur ma proposition, le délai dans lequel le bénéficiaire doit confirmer l'existence du pacte et son intention de sa prévaloir, dire que la commission d'ailleurs entre délais raisonnables, délais de moi vous certains avaient également dit que ce délai était encore éventuellement trop long, ce délai, bon nous semble suffisant pour confirmer l'existence d'un Pack de préférence et accomplir les diligences nécessaires préalables à la décision de s'en prévaloir, pourquoi encore, la commission a-t-elle fixé ce délai, ce qui pourrait vite. T. et effectivement des contentieux attiré votre attention peut-être à Pékin, peu de malice sur le fait que, devant la cour d'appel lorsque la plante conclu : certes, il peut pas faire de demande nouvelles mais il peut évoquer des moyens nouveaux et que celui qui répond à un délai qui me semble bien. Préfixe de 2 mois ou en tout cas peu rallonge pour quelques fois répondent à des questions techniques extrêmement précises, je ne vois donc pas d'ailleurs pourquoi, dans cette hypothèse-là le la personne qui se voit interrogé ne pourrait pas répondent dans le délai de moi là encore il s'agit, discussions qui peuvent qui peuvent éventuellement s'éterniser la commission des Lois, essayer de trouver un système intermédiaire pour éviter des coûts tentation. Donc j'en conclus bien du Bruxelles défavorable, monsieur le rapporteur, donc est-ce qu'il y a des explications de vote Monsieur Bigot. Oui, merci de ce débat en séance, Madame la Ministre Monsieur rapporteur j'avoue qu'en commission, j'avais fait l'observation disons de mois c'est un peu court et finalement un ministre, je pense que vous avez raison de dire que le pacte de préférence le le va dire à celui qui bénéficie du parc du pacte prononcez-vous, il doit lui donner un délai si le délai considéré par celui qui doit se prononcer comme déraisonnable il invoquera ultérieurement, justice, donc je pense que cette liberté laissée aux partis et suffisant parce que le délai de 2 mois, parfois risque d'être trop long, je pense qu'il sera rarement trop court mais qu'il faut qu'il vaut mieux en fait effectivement voir cette souplesse, c'est vrai que ça peut ouvrir sur ce contentieux mais finalement celui qui interroge le le tiers bénéficiaires du Pacte a tout intérêt aussi à ne pas rester trop longtemps dans l'incertitude et à lui convenir avec lui du délai raisonnable qu'il lui faudra pour répondre donc je pense que cette souplesse et mieux pour la pratique et je propose que, pour notre groupe, nous suivions, madame la ministre, votre amendement.

Très bien, pas d'autres explications, cette fois-ci, donc je soumis au vote, je rappelle la Commission défavorable gouvernement évidemment favorable qui est pour cet amendement.

Qui contre. Il est donc approuvé. Article 5, nous allons examiner l'amendement 4 rectifier bis Madame Mellow. Merci madame la présidente. Il s'agit de de du nouvel article 1132 du code civil qui a introduit l'erreur de droit jusqu'à présent inconnue en droit français, en consacrant l'erreur de droit, l'article 1132 nouveaux du code civil, porte atteinte à la règle selon laquelle nul n'est censé ignorer la loi, le risque est que le justiciable puisse faire échec à l'application de dispositions supplétives ou impératif de droit objectif normalement applicable au contrat en invoquant une erreur de droit et porte ainsi atteinte à la force obligatoire des contrats autres, les rares de droit n'est pas définie, il pourrait tout aussi bien s'agir d'une erreur sur la signification d'une règle de droit positif que d'une erreur sur la porte et où les conséquences des stipulations contractuelles il convient dès lors de supprimer toute référence à l'erreur de droit aussi au sein de l'article 1132 nouveaux du code civil, merci.

pour autant, rien n'est dramatique puisque l'ordonnance ne fait que consacrer la jurisprudence sur ce point, et l'article 1132 du code civil est clair : l'erreur inexcusable non porte pas nullité du contrat, elle est portée sur une qualité essentielle de la prestation ou de la personne, c'est la raison pour laquelle la commission des lois, a précisé l'interprétation qu'il convenait de faire de cet article sans pour autant le modifier dans les conditions que chez expliqué tout à l'heure dans le cadre de la de la méthode que j'ai expliqué tout à l'heure, il n'est en effet nullement question d'élargir leurs missions de l'erreur de droit, en permettant un compte un contractant de prétendre qu'il s'est mépris sur la portée d'un texte légal d'une jurisprudence ou même de son engagement contractuel en effet si la jurisprudence admet l'erreur de droit, c'est à ce titre qu'il est légalement consacré et l'a toujours fait une application mesurée en la refusant lorsqu'elle portaient par exemple sur une décision judiciaire s'était rendu pour d'autres partis ou sur les effets que le contrat doit produire, donc, au regard de l'interprétation Express sur laquelle on attire l'attention des magistrats et des juristes qui ont appliqué cette article. J'ai aimé la commission émet un avis défavorable, mais je vous dis toujours loisible de retirer votre amendement. Madame la garde des Sceaux, l'avis du gouvernement. Même avis que monsieur le rapporteur. rapporteur. Madame vous retirer. Madame la présidente, je vais le retirer. Nous passons donc à l'amendement numéro 16 heures, présenté par le gouvernement.

et d'en exclure l'estimation de la valeur de la prestation, la réticence de l'ogive consiste à retenir sciemment une information dont on sait le caractère déterminant pour l'autre partie, et qui, si elle avait été connue de cette dernière, l'aurait amené à ne pas contracter ou à contracter. à des conditions substantiellement différente untel comportements contraires au devoir de bonne foi, contractuels et sanctionnées par la nullité du contrat la rédaction adoptée par la commission des lois subordonne cette sanction à la violation préalable d'un devoir légal d'information, or il nous semble que Le Devoir précontractuel d'information instaurer comme nous l'avons vu tout à l'heure à l'article 1112 Tiret est strictement encadrée il n'est due que si l'ignorance de l'autre partie était légitime ou si elle pouvait en raison des circonstances, faire une confiance particulière à son co-contractant la réticence de Lozi qui implique une intention de trop. P. ne doit pas être assujettis aux mêmes limites, ce n'est pas la même chose, la mauvaise foi, implique que le Dol doit en effet être sanctionné plus largement. Plus réellement que la seule négligence dans la délivrance d'informations, c'est pourquoi je vous invite au rétablissement du texte initial, toutefois, afin de ne pas pénaliser le commerce, je vous propose que le silence même intentionnelle sur l'estimation de la valeur de la prestation soit exclu de la sanction comme 2 du Dol, comme il est exclu du devoir d'information. Rapporteur pour la commission. L'amendement proposé par le gouvernement, donc vise à exclure l'estimation de la valeur de la prestation du Champ d'application de la rive distance de Lozi afin de consacrer la jurisprudence bien connu au moins des professionnels dites Bâle du s'si je suis favorable à la à la consécration de cette jurisprudence, j'estime que cet amendement ne résout pas toutes les difficultés soulevées par l'incohérence des champs d'application respectif des articles on 112 et 137 137 du code civil, que la commission des lois entendu résoudre ces difficultés ont d'ailleurs été évoquée par la quasi-unanimité des personnes que j'ai entendu lors des auditions, or avec la rédaction, telle que proposée par l'amendement des incohérences, à mon sens subsisteraient certaines informations non visés par l'obligation d'information de l'article 112 1 du code civil, car elles ne sont pas déterminantes au sens de cet article, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de lien Direct et nécessaire avec le contenu du contrat, la qualité des partis pourrait en revanche être considérée comme déterminante au sens de l'article 137 du même code en fait la réflexion de la commission. Fait sur le les 2 textes pour les rendre plus plus plus homogène. De surcroît, le Dol implique une dissimulation intentionnelle, or il semble que la dissimulation d'une information est par nature intentionnel, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le Champ d'une obligation d'information, ce sont les raisons pour lesquelles je souhaite le maintien de la rédaction de la commission des lois, qui permet de subordonner la nullité pourquoi ici réticences Delaisi aux hypothèses dans lesquelles une obligation d'information préalable existe, je précise, en outre, ce qui n'est pas un élément anodin que la rédaction de la commission des lois, reprend exactement celle qui était proposées par l'avant-projet d'ordonnance qui avaient été publiés par la chancellerie en 2015 et soumis à la consultation publique en quelque sorte, je pense que le premier éléments qui avait été donc publié la première réflexions de la chancellerie n'aurait pas mérité que la consultation publique la modifier. Explications de vote Monsieur Bigot. Oui, le débat technique prouve bien que finalement on aurait dû avoir un débat complet sur le texte, mais goût de l'amendement du gouvernement et, aussi, ne l'oublions pas de supprimer ce que vous modifiez, monsieur le rapporteur sur la notion de de réticences de l'audit, vous mettez dans votre article que l'information doit uniquement porté sur l'obligation faite à l'autre partie, conformément à la loi, or ce qui est important, c'est que dès lors que l'une des parties, c'est que l'information était déterminante du consentement de l'autre, elle devait fournir cette information et j'en réfère là ce que disait alors dans mon intervention liminaire, c'est la notion de bonne foi qui doit primer cette notion, elle remonte Portalis à d'autres et dans votre rédaction cette bonne foi disparaît parce qu'effectivement, il faut simplement soit prévue par la loi, or la loi ne prévoit pas tout en matière d'information, loin s'en faut, et donc effectivement l'amendement du gouvernement paraît meilleure et c'est pas par hasard que l'ordonnance dans sa mouture définitive n'est pas dans le la même veine que la première il y a une amélioration entre les 2 premiers textes et moi je préfère le 2ème texte rétabli par le gouvernement avec la précision, Madame la Ministre, que vous apportez, donc je propose à mon groupe de voter l'amendement du gouvernement. la bonne foi de toute façon il couvre tous les domaines du taxer tout le domaine de la réforme donc, en toute hypothèse, la bonne foi n'est pas exclu de l'application et de l'interprétation de ce texte. de ce texte. Les explications de vote non, je vais donc soumettre, voici l'amendement numéro 16 avec un avis défavorable de la commission évidemment une avis favorable du gouvernement. Qui est pour.

résultant de la dissimulation intentionnelle par l'un des comptes co-contractants d'une information dont il c'est le caractère déterminant pour l'autre partie, autrement dit la réinvestissant ce de Lozi d'une telle omission donne la possibilité à la partie qui se prétend victime d'une réticence de logique d'obtenir la nullité d'un contrat, alors même qu'elle aurait failli à son devoir de se renseigner l'excuse automatique de l'erreur, provoquée par une réticence Deleuze Yves risquant d'exonérer le co-contractants de tout devoir de se renseigner, il convient que l'article 1139 nouveaux du code civil précise que l'erreur résine tendent une réticence Deleuze Yves n'est Xtube Kusama que si la victime ignore légitimement l'information qui lui a été dissimulé intentionnellement. Avis du rapporteur. où la rédaction adoptée à l'article 1137 subordonne la nullité pour réticences de l'Asie vos hypothèses dans lesquelles une obligation légale d'information existe, il n'est aucunement besoin de modifier, article 1139 du code civil afin de transposer un devoir d'information alors qu'il est déjà prévue à l'article 112 1 du même code donc le l'objet de votre amendement me paraît assez avec beaucoup de précision. Satisfait déjà dans le texte et je vous suggère de le retirer, sinon ce serait un avis défavorable. Le gouvernement madame la garde des Sceaux, même avis mais méfiez-vous Madame Mellow vous maintenez votre amendement. Non, non, madame la présidente, je me retire, merci pour ces explications. Merci madame, nous passons, ensuite à l'examen de 2 amendements identiques, l'amendement numéro 1 présentée par Monsieur Collombat et l'amendement numéro 15 présenté par le gouvernement Monsieur Collombat. notre reporter et une notre commission ont cru bon de préciser la notion de limiter la notion de dépendance à la dépendance économique. nous pensons qu'il vaut mieux garder le terme l'acception du terme dans sa vie dans sa généralité et couvrir la totalité des situations de de dépendance, alors on m'objecte que c'est déjà fait. Quelque part, dans telle dans telle autre, enfin

Madame la garde des Sceaux pour défendre crânement. Celui du gouvernement oui. Donc, je suis favorable à l'amendement de monsieur Collombat qui reprend effectivement l'amendement du gouvernement. Qui est identique, pardon. Non mais reprend, c'est bien aussi l'article 1143 du Code civil et l'une des innovations essentielles de l'ordonnance du 10 février il assimile à une violence l'abus de dépendance dans laquelle se trouve le co-contractants, ce que la jurisprudence de la Cour de cassation a admis dans plusieurs arrêts récents et que la doctrine et les praticiens qualifient de violence économique : le texte adopté par le gouvernement se veut néanmoins délibérément plus large puisqu'il n'est pas circonscrit à la seule dépendance économique toutes les hypothèses de dépendance sont visés, ce qui permet une protection des personnes vulnérables, et non pas seulement des entreprises dans le rapport entre elles, ce choix est d'ailleurs conforme au terme de l'habilitation qui a été accordé par le Parlement au gouvernement puisque cette habilitation autorisé le gouvernement à introduire des dispositions, je cite, permettant de sanctionner le comportement d'une partie qui abusent de la situation de faiblesse de l'autre, il pourrait donc s'agir d'une situation de dépendance sociale ou psychologique, ce qui pourrait permettre de sanctionner un abus commis par exemple à l'encontre de personnes âgées dépendantes d'un point de vue affectif, voire psychologique à ce titre, les dispositions qui sanctionne l'abus de faiblesse dans le code de la consommation dans le code pénal ne sont pas comparables puisqu'elles édictent des sanctions pénales sans prévoir l'annulation du contrat conclu et que tant leur Champ d'application que leurs conditions de mise en oeuvre diffère de ceux de l'article 1143 en effet, la faiblesse et l'ignorance visés au code de la consommation ne sont pas synonymes de dépendance et ces dispositions ne s'appliquent. Que dans les Que dans les relations entre professionnels et consommateurs quant aux dispositions pénales, elle ne concerne que les abus à l'encontre des mineurs ou de personnes, d'une particulière vulnérabilité en raison de leur âge, de leur maladie ou encore d'une infirmité si j'entends bien entendu les inquiétudes légitimes exprimées sur l'appréhension des notions d'abus et de dépendance, il me semble que le texte de l'ordonnance prend le soin de poser des conditions objectives tenant d'une part à l'existence d'un Avantage manifestement excessive et d'autre part à ce que la dépendance est une notion elle-même objectives qui ne tient pas uniquement aux qualités de la victime de l'abus, comme dans les textes du code de la consommation et du code pénal, mais également aux circonstances de la conclusion du contrat en cause, il est indispensable, me semble-t-il, doter notre notre droit des contrats d'un outil de contrôle des abus, des situations de faiblesse en dehors des seuls régimes pénaux spéciaux, je vous demande, en conséquence, mesdames et messieurs les sénateurs, de bien vouloir rétablir le texte de l'ordonnance dans son intégrité. L'avis de la Commission, monsieur rapporteur président.

la motivation de de vos amendements. Pourquoi je ne la partage pas parce que les exemples que vous prenez sont déjà traitées par par la le régime de protection légale des incapables, permet de garantir une protection juridique pour les personnes concernées en état de faiblesse, de même le code de la consommation permet la sanction de l'abus de faiblesse ou d'ignorance, enfin pour les abus commis à l'égard de personnes âgées en situation de dépendance illettrés ou sous l'emprise d'une secte qui sont évoqués dans votre amendement madame la garde des Sceaux, l'article 223 15 du code pénal réprime déjà l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'un mineur ou d'une personne d'une vue la vérité particulière qui l'a conduit à un atout, une abstention qui lui sont gravement préjudiciable si imaginons alors ces textes déjà apporte la protection qu'est qui est attendu, imaginons qu'il a une sanction pénale, comment pourrait-on imaginer que le juge pénal ne prononce pas la nullité de la résolution du contrat alors qu'il y a eu la carte qui a été caractérisée soit un vice du consentement soit une fraude. Je pense que sur ce point, vous pouvez vous pouvez tracer rassuré, en revanche, en revanche, si nous gardons le terme dépendance sans précision nous introduisons tout de même une un caractère très imprécis et incertain de cette notion, qui ne serait pas qualifié et qui me paraît très posé problème alors pourquoi dépendance économique parce que c'est une notion qui a parfaitement été déjà encadré par la jurisprudence et je pense très honnête. Non mais je veux bien qu'on puisse encore en discuter au cours de de la navette. Je pense très honnêtement que toutes les hypothèses que vous pouvez imaginer sur l'état de dépendance sont déjà couvertes par tous les autres aspects du droit et qu'il n'y a pas lieu dans ce domaine très général d'introduire une notion qui serait à mon sens imprécises, c'est sous bénéfice de ces observations que vous considérez, je pense comme très mesuré que j'aime être un avis défavorable.

devaient être censées être parfaitement autonome dans leur volonté capable petit à petit, on s'est rendu compte quand même au bout de siècle qu'il y avait des gens qui étaient dominés et que il fallait trouver des moyens d'annuler le contrat en considérant que le vice du consentement AT obtenu par la violence ou sur d'autres motifs, alors certes, il y a eu toute une série de combat pour obtenir l'abus de faiblesse sur les personnes vulnérables et âgé, il a mis du temps à faire, à le possibilité de remettre en cause un acte pris par quelqu'un qui était incapable, on a dû inventer la sauvegarde de justice etc, donc ce n'est pas aussi simple que ça, ce que le texte de loi prévoit, c'est effectivement l'état de dépendance dans lequel se trouve son contractant et grâce à l'auquel on obtient un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et on en tire un Avantage manifestement excessif pour celui qui l'obtient, on est là dans une protection des personnes vulnérables, le fait de préciser dépendance économique tend à réduire la portée du texte, alors que là, il était l'argile, moi, mes chers collègues, je vous rappellerai que ce texte il date d'octobre, le 2 février même 2016 donc sous en gouvernement qui était franchement à gauche et que, aujourd'hui, on sent bien qu'il y a un courant encore libéral et de droite qui est plutôt restrictif et donc nous allons suivre l'amendement de monsieur Colomba et du gouvernement parce que Madame la Ministre, pour une fois, il est plutôt de gauche comme de droite.

bien là qu'est-ce que c'est que une dépendance économique, une personne qui a pas mal d'argent mais qui est trop âgé pour pouvoir véritablement être considérés comme autonomes. autonomes. Dans quelle situation. Et pour une dépendance économique, c'est simplement que qu'elle a pas les les moyens véritablement de prendre la la bonne décision, alors oui, oui, on va les chercher dans telles code on aura toujours la solution etc mais qu'est-ce qu'on fait là.

madame la présidente, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs, il me semble effectivement que là nous sommes sur une je dirais un une divergence apporter un peu politique

que le juge pénal dans les autres dispositions, vous avez évoqué, ainsi que je l'ai dit tout à l'heure, n'a pas exactement les mêmes pouvoirs que ce qui est ici proposé, il n'a pas dû n'est pas en capacité de prononcer l'annulation du contrat et donc si vous voulez, je crois qu'il y a là réellement des dimensions différentes, et moi je, vraiment, je souhaiterais que nous puissions revenir à l'écriture initiale du texte. Monsieur le rapporteur, je vous signale qu'il faut être assez brève parce qu'on va devoir suspendre la séance. Si vous promettent de l'être, rassurez-vous, chers collègues, j'ai parfaitement vu vu vulve le problème : il ne s'agit pas, j'allais même dire de d'introduire quelques notions même ma légère fragmentation politique dans la rédaction de ce texte mais nous avons, nous avons des, des, des éléments légaux de protection des personnes qui sont en état de dépendance, puis nous avons une autre notion tout en autre kyrielle de possibilités, c'est le vice du consentement qui les protège également, c'est la raison pour laquelle, moi j'avais pensé que je ne devais aider je ne venais pas particulièrement oublieux des personnes dépendantes en limitant uniquement la à la dépendance économique qui est une notion jurisprudentielle et comme je veux montrer que le Sénat irresponsable et qu'il est capable de débat, ce que je propose, sous réserve que l'on admette d'à peu près de modifier, de réfléchir à cette définition afin qu'elles deviennent plus précises, hé bien c'est de rechercher

parfait donc bien amendements avis défavorable sur les 2 s'amendement de la commission et avis favorable du gouvernement il y a plus d'explications de vote soumet donc à votre vote qui, pour ces 2 amendements identiques. Qui est contre. Les amendements ne sont donc pas adoptée, nous allons donc soumettre à votre à votre vote, l'article 5 qui est pas d'explication de vote qui est pour l'article 5. Qui est contre. L'article 5 et donc adopté je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 16 heures 45 pour les les questions d'actualité au gouvernement, la séance est suspendue.

La séance est reprise. Monsieur le 1er Ministre Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, notre ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement, nous sommes retransmis en Direct sur Public Sénat sur le site internet sur Facebook, je rappelle à chacun, à la fois le respect du temps j'ai insisté avant de passer aux mesures Commercy tive donc que chacun soit respectueux les uns des autres et naturellement le respect qu'on se doit mutuellement la parole est maintenant notre collègue Brigitte Lherbier pour le groupe, les républicains. Monsieur le Monsieur le Ministre, monsieur le 1er ministre Monsieur le ministre de l'Intérieur, sur le site internet de notre ministre de votre ministère, on peut lire, je cite : l'étranger qui souhaite venir en France, doit-il être autorisé. Présent sur le territoire national centilitres l'étranger est alors en situation irrégulière, il s'agit d'un rappel de la loi française votée par le Parlement, force est de constater que la loi, comme c'est malheureusement trop souvent le cas n'est pas peu appliquées concernant la terrible affaire de Marseille où 2 jeunes filles ont été sauvagement tués l'assassin était un clandestin et avait commis des délits à répétition, on estime à plusieurs centaines de milliers le nombre d'étrangers qui séjournent illégalement dans notre pays, lors de son intervention télévisée dimanche soir le président de la République a tenu des propos fermes contre l'immigration illégale, il a promis l'expulsion de tous les étrangers en situation irrégulière ayant commis un délit, quel qu'il soit. Sa proposition mérite des éclaircissements : s'agit-il pour le président de la République de limiter les expulsions clandestins qui auraient commis un délit, la langue du président de la République a-t-elle fourché à-t-il cultiver une savante ambiguïté ou ça ou avait-il bien à l'esprit une vision restrictive des reconduites à la frontière, c'était l'Erika j'attire votre attention, monsieur le Monsieur les ministres sur le fait que la loi française prévoit l'expulsion de tous les clandestins qui ait commis ou non Adèle et que de limiter l'expulsion à ceux qui auraient commis un délit redevient redevient reviendrait à donner un droit de séjour. En France, aux étrangers illégaux, merci monsieur le ministre de l'intérieur de nous éclairer sur les intentions précises du président de la République et en même temps de lever toute ambiguïté sur ses propos. Merci pour vous répondre. La parole est à Madame Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, vous avez la parole. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Brigitte Lherbier, en effet, les services de l'État doivent être pleinement mobilisé pour éloigner les étrangers en situation irrégulière qui présentent une menace pour l'ordre public, vous l'avez rappelé le président de la République a confirmé cette orientation prioritaire et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur a, dès le 10 réécrit au préfet, dans une circulaire pour leur préciser bien sûr que l'ordre public devait être respecté et que les sortants de prison devait faire l'objet d'une attention prioritaire notre droit, nous permet de les éloigner, vous avez raison, en prenant à leur encontre une OQTF sans délai de départs volontaires, mais aussi en permettant de les placer en rétention s'ils présentent un risque de fuite. Pour les sortants de prison, une meilleure articulation doit être recherchée avec les établissements pénitentiaires pour mieux anticiper les éloignements durant la phase d'incarcération, c'est absolument certain, par ailleurs, pour faciliter l'identification des personnes interpellées, un système biométrique relié au fichier de gestion des dossiers des étrangers sera déployée dans les prochains mois, il permettra la consultation du fichier à partir des empreintes digitales de la personne, dans le même objectif, les forces de l'ordre seront dotés, en 2018 d'équipements permettant de prendre les empreintes digitales sur place et de consulter les fichiers de façon mobile madame la sénatrice, comme vous le voyez bien sûr, il y a une politique ferme à cet égard, et par ailleurs bien sûr ceci n'empêche pas d'accueillir. Comme c'est la tradition dans notre pays, les réfugiés qui chilienne demander l'asile dans notre pays, car ils sont menacés dans leur propre pays, bien évidemment, je vous remercie. la parole est à Madame Élisabeth Doineau. Pour le groupe de l'Union centriste avait la parole pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président, chers collègues, cette question s'adresse à Madame la ministre de la Justice, Garde des Sceaux, mais elle pourrait s'adresser aussi au 1er ministre comme au ministère de l'Intérieur, comme au ministère des Affaires étrangères ou des affaires sociales, la question étant très large, le 5 septembre dernier le président de la République a demandé au gouvernement des propositions pour revoir l'accueil et l'accompagnement des mineurs non accompagnés, il précisait que la réponse actuelle n'est pas satisfaisante et qu'elle représente une charge croissante pour les départements dans le rapport d'information que j'ai présenté dernièrement avec mon ancien collègue Jean-Pierre Godefroy nous annoncions une explosion des prises en charge de 13000 situations à la fin décembre 2016, nous passerons à 25000 à la fin de l'année, tous les départements sont touchés, avec des records jamais atteints, les agents des départements sont dépassés, voire en berne Out professionnels parce que nous ne sommes plus dans le Champ de nos compétences, cela va jusqu'à mettre en danger notre mission historique de protection de l'enfance 1er problème les berges ment aujourd'hui, nous observons une embolie de toutes nos structures d'accueil malgré leur diversité et leur nombre 2ème problème : l'évaluation de la minorité nos services sont totalement accaparé et décourager difficulté d'authentifier les documents administratifs, quand il y en a, avec des appréciations variable selon les préfectures, difficultés de bénéficier des services d'interprètes, parce que trop rares difficultés d'analyser les parcours migratoire chaotique de ces jeunes qui mériterait l'appréciation des services de la police aux frontières 3ème problème l'accompagnement que leur proposer comme formation sinon l'apprentissage, mais là encore, nouveau parcours du combattant, je pourrais continuer ainsi pendant longtemps parce qu'il faudrait aussi parler des multi traumatismes ressentis par ces jeunes, il faudrait aussi parler des Liens avec les parquets et les cours de justice qui sont également dépassées par le nombre et des recours, portés par les avocats Vaudois j'Annonciation, c'est une question qui relève des flux migratoires et c'est à l'État de prendre ses responsabilités dans ce domaine, les conseils départementaux sont dans l'attente de mesures concrètes. Pour vous répondre, la parole est Avram, le garde des Sceaux, madame Belloubet. Monsieur le Président, Madame la sénatrice de nos mesdames et messieurs les sénateurs, effectivement, Madame la sénatrice, vous avez raison de souligner témoignent de oui oui je vous vois vous avez énoncé des chiffres qui témoignent de l'urgence de l'acide. Création, nous en sommes pleinement conscient, je dois vous dire qu'avec ma collègue Agnès Buzyn, nous avons tenu le 15 septembre dernier un comité de pilotage

qui est destiné à prendre en charge l'évaluation et la mise à l'abri qui est assumé par les départements, nous avons également réaffirmé que l'État tiendrait ses engagements qui consistent à rembourser au département 30 pourcent du du coût qui correspond à la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance menaces supplémentaires, ceci pour l'année passée, mais nous savons, et vous l'avez rappelé à juste titre qu'il y a de grandes difficultés, notamment concernant la phase d'évaluation et de mise à l'abri de ces jeunes, nous savons pertinemment que des jeunes qui sont déclarés majeurs dans un département se représente dans un autre département, pour tenter de faire connaître leur minorité, donc nous devons établir des soutiers qui nous permettent d'éviter cela, nous devons harmoniser les procédures d'évaluation pour qu'il n'y a pas difficulté avec les parquets et ensuite, bien entendu, il y aura la prise en charge de ces jeunes lorsque leur minorité aura été reconnu monsieur le 1er ministre qui se rendra vendredi à l'assemblée départementale, aura à cette occasion, la possibilité de vous faire je crois que des annonces d'un plan d'action très concret. Si Madame la Ministre Monsieur notre collègue Frédéric Marchand pour le groupe de la République en marche. Monsieur le président, Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de la cohésion des territoires, monsieur le ministre, la politique de la ville est né il y a 40 ans, avec les premières opérations Habitat et vie sociale prémices de la politique de la ville et de sa méthode, malgré l'engagement des acteurs sur le terrain et des progrès réalisés en matière de cohésion sociale, de cadre de vie, de renouvellement urbain et d'emplois, le regard porté sur les quartiers populaires, reste aujourd'hui encore trop souvent négatifs et trop souvent stéréotypé, vous le savez, les habitants de ces quartiers ne veulent pas être assigné à résidence, bien au contraire, il revendique de la dignité de la considération et bien évidemment du travail maire pour encore quelques jours d'une commune dans la métropole lilloise dont 2 quartiers sont inscrits en politique de la ville depuis le 1er janvier 2015, je suis comme tous les élus, conscients de la nécessité d'engager une nouvelle étape pour tenir cette belle promesse républicaine qui nous est chère : l'égalité des territoires, monsieur le Ministre, au-delà des premières décisions prise sur cette grande cause nationale je pense ici notamment aux classes dédoublées de CP en REP plus et dont chacun salue en cette rentrée scolaire, la pertinence, pouvez-vous nous indiquer les mesures qui seront Mist en oeuvre dans les prochains mois pour conforter ses territoires urbains en souffrance dans des domaines aussi essentiels du quotidien que sont le logement, l'emploi, l'éducation ou bien encore la sécurité, je vous remercie. Pour et prendre la parole est 26 Jacques Mézard. Ministre de la cohésion des territoires, vous avez la parole Monsieur le Ministre. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, marchand, j'entends le message des élus locaux, des maires, relatif à la politique de la ville, nous connaissons la fragilité de nombres de ces quartiers où l'avait rappelé ça fait 40 ans que cette politique de la ville a été lancée avec des roues avec débat si la réussite avait été totale il y aurait plus politique de la ville, nous sommes face à des situations très diverses, d'ailleurs, et ce que souhaitent, ce que souhaitent nos concitoyens, les habitants de ces quartiers, les élus se sont d'avoir assez d'avoir les mêmes droits, les mêmes chances, ça s'appelle le droit commun ce qu'ils veulent, alors je voulais d'abord préciser les choses en ce qui concerne les questions budgétaires sur la 1ère étape de l'engagement que nous avons pris autour du 1er ministre c'est la mort de reconduire le budget de politique de la ville en 2018 430 millions d'euros et pour les années suivantes aussi d'avoir 150 millions d'euros sur la DPJ de mètres 90 millions d'euros supplémentaires sur la DSU, voilà une réalité financière budgétaire ensuite et vous l'avez dit avoir une politique forte en ce qui concerne l'éducation. Où il y a beaucoup à faire et ce qui a été mis en place avec 2500 classes dédoublées dans ces quartiers, parce que ce sont surtout les réseaux d'éducation prioritaire plus et qui ont été visés, je pense qu'on voit déjà que c'est une politique extrêmement volontariste et est très forte, nous allons aussi mettre en place bientôt des emplois francs sur ces quartiers, politique de la ville et puis vous avez parlé de sécurité parce que la sécurité à l'est essentiel dans ces quartiers, il faut vraiment qu'il y a une police de proximité, il y a des efforts considérables à faire, car nous avons à lutter contre le communautarisme, tous ensemble, parce que si la République recule dans ces quartiers, il y en a d'autres qui vont prendre sa place et qui sont déjà au travail et ça, c'est un enjeu tout à fait fondamental et tout à fait prioritaire et j'entends que nous menions une politique interministérielle car nous avons besoin d'avoir sur tous les sujets politiques très fort, voilà ce que je voulais vous préciser, Monsieur le Sénateur, dans le cas de ce dossier. Merci, monsieur Dominique. Ce marchand est-ce que vous souhaitez répliqué Monsieur ce que les fans Artano mon cher collègue, pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, de l'Outre-mer voulons serait jeudi à Saint-Pierre-et-Miquelon, les assises de l'Outre-mer, voulue par le président de la République, j'espère qu'elle ne connaîtront pas le triste succès des états généraux, je formule donc le voeu sincère qu'elle soit un véritable succès pour la République depuis 8 ans sur mon territoire, les élus du conseil territorial réconcilie la politique et la société civile par une démocratie participative permanente et renforcée, je me félicite donc de votre initiative ambitieuse mais en posant comme postulat que les assises permettront quelque part de réinventer les outre-mer, certains pensent déjà que les élus ultramarins n'ont rien fait pourtant nos territoires sont en mouvement. à Saint-Pierre-et-Miquelon, en 2009 nous avons au travers d'une démarche innovante du territoire adopter un schéma développement économique sur 20 ans. Ce schéma, développement économique, a reçu le soutien de l'Union européenne. Nous avons adopté avec l'État, tout récemment, en 2015 no 38 mesures concrètes qui vont occuper le territoire pour les 5 ans qui viennent, en mars 2017, c'est cette démarche innovante qui nous a permis de convaincre 70 pourcent de de la population sur ce plan, développement économique, madame la ministre, vous avez évoqué que ces assises seront finalement la feuille de route de les politiques publiques en outre-mer pour le quinquennat il ne faut pas vendre du rêve aux concitoyens qui attendent des projets concrets. L'État respectera-t-il la légitimité électorale des programmes de développement économique en cours. Comment ne pas craindre une cacophonie ou un mélange des genres entre la tenue des assises l'élaboration concomitante des projets, État, collectivités, au pluriel et le plan de convergence de la loi Égalité réelle, ce sont 3 documents différents avec des vocations différentes comment organiser vous cette articulation,

Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, comme vous le savez, et comme vous l'avez dit, le président de la République a souhaité que dans sa compagne électorale les Assises des Outre-mer soit organisé de début de ce quinquennat l'objectif des assises, c'est bien sûr de construire des politiques innovantes de réinventer de nouveaux outils, tout en évaluant, bien sûr, ce qui existe pour construire notre parcours commun sur ce quinquennat tous les sujets peuvent être abordés et chaque territoire est libre de choisir ses sujets Mayotte par exemple choisi la question et on peut le comprendre, c'est une priorité de la sécurité, la Calédonie souhaite évoquer la question de de la jeunesse, Saint-Pierre-et-Miquelon, mais effectivement un certain nombre de priorités avec les élus locaux, mais aussi avec la société civile et c'est très important dans ce cadre, il y a également une plateforme numérique, qui a été lancé et qui permettra que l'ensemble des citoyens des territoires d'outre-mer puisse s'exprimer, ce qui le plus souvent non pas la parole, et on souhaite effectivement renouer ce lien avec eux alors vous interroger Monsieur le Sénateur, sur l'issue des assises de leur traduction législative ou encore leurs Liens avec les autres exercice démocratique qui ont lieu sur le territoire alors rassurez-vous, l'idée n'est pas de tout oublier, mais bien de remettre remettre en perspective, un certain nombre de projets de territoire et surtout d'apporter des réponses en matière d'outils d'outils précis de projet précis à ce que vous souhaitez mettre en place sur les les territoires, nous voulons créer un véritable écosystème économique pour aider le développement des territoires, mais bien sûr de pouvoir accompagner aussi l'ensemble des projets sociaux alors prenons tous on à notre avenir et participants à ces assises à tous les niveaux pour apporter une réponse à ceux qui l'attendent une réponse efficace efficace une réponse qui se veut co-construite et je crois que c'est une méthode que qu'il m'est cher, c'est-à-dire comment co-construire ces défis communs que nous avons et comment surtout répondre à l'ensemble des exigences et des défis que doivent relever aujourd'hui les territoires d'outre- mer, merci. Merci mon ami Monsieur Hart, alors vous avez dit seconde. Merci monsieur le président, n'oubliez pas que les initiatives viennent des territoires, l'innovation est déjà présente les programmes existent, il suffit simplement que le gouvernement les respecte. Merci, la parole est. Notre collègue Pascal Savoldelli pour le groupe communiste républicain et citoyen et écologiste avait la parole. Monsieur le président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, faute de ministre du Logement, cette question va donc s'adresser au ministre de la cohésion des territoires. Les déclarations du président dimanche ont suscité une profonde indignation. Il a ainsi déclaré et je le cite dans le monde HLM il y a des réserves, on le sait depuis des décennies, il y a des acteurs qui ont beaucoup d'argent. Il poursuit dans le monde HLM il y a des organismes qui ont de l'argent et qui ne le dépensent plus on construit une forme de rente. Je vous pose la question : quel est le montant de cette trempe, Monsieur le Ministre, avez-vous des chiffres avancés après ces graves accusations. Rappelons que les moyens des offices Comolli oblige la loi, son rêve réinvestis dans l'économie réelle au service des locataires dans la construction, la réhabilitation et jamais distribués sous forme de dividendes après la manifestation de samedi pour le maintien des APL, plusieurs rassemblements se tiennent aujourd'hui pour la défense de l'habitat social des locataires et des personnels des bailleurs sociaux. J'entends dire souvent de la part de ministres, je cite, que la rue ne fait pas loi mais Monsieur le Ministre, la rue, c'est aussi la République sociale est inscrite dans notre constitution, alors vous devez répondre aux questions posées, les 3,2 milliards d'euros pris sur 2 ans au logement social et aux bailleurs, à quoi va-t-il servir est cela que vous allez chercher le financement des nouveaux cadeau fait aux riches qui coûteront la bagatelle de 4 milliards d'euros.

plus de 40 milliards d'euros consacrés par l'État, au logement et encore 4 millions de mal-logés, il y a là une responsabilité collective qui ne date pas d'aujourd'hui, votre question, je peux la comprendre, je respecte tout à fait les sensibilités diverses et l'expression aussi de la rue et aussi, vous savez, je suis allé au congrès de l'USH, j'ai passé un bon moment, comme vous le savez, mais c'est la vie c'est la vie démocratique, simplement je crois que nous avons une responsabilité collective et d'ailleurs le Sénat apporte sa contribution au niveau de du travail qui est fait depuis des années, ici sur le logement, et nous en tiendrons le plus grand compte simplement vous dire que. Je ne vais pas m'abriter derrière les rapports de la Cour des comptes, je sais ce que d'aucuns ici peuvent en penser, y compris dans votre groupe, mais quand même, j'ai souvent entendu ici parler des dodus dormants, ça veut pas dire que toutes les structures HLM sont dans la difficulté mais ça veut dire ça veut dire très simplement qu'il y a une grande diversité et qu'il y a nécessité de restructuration qu'il y a nécessité de mutualisation m'apporter celle de du secrétaire d'État a toujours été ouverte pour le dialogue avec les bailleurs sociaux, elle continuera à l'être, nous avons fait monsieur le 1er ministre a fait des propositions de compensation qui ne sont pas neutres ce dialogue, je vais avec l'ensemble du gouvernement, le poursuivre et je suis sûr que nous allons trouver des solutions, c'est le cas de le dire constructive. Monsieur le Ministre, chers collègues, dont 27 secondes. Vous apprécierez la réponse à la question d'abord Monsieur le mini-je vous rappelle, vous devez aux organismes HLM, c'est la dette de l'État 2 milliards d'euros, donc tout ça, vous avez pas répondu y compris pourquoi vous faisiez s'économie par rapport, moi je le pense, par rapport à l'ISF, donc ça s'appelle une politique de classe et c'est comme ça, donc, permettez-moi d'adopter une phrase de Jules Renard, Monsieur le Ministre, si on doit fêter votre politique du logement, la plus grande pièce 500 la salle d'attente. La parole est maintenant notre collègue il Yannick Vaugrenard, pour le groupe socialiste et républicain, vous avez la parole. mesdames, messieurs, mes chers collègues, ma question s'adresse au 1er ministre la journée mondiale du refus de la misère et précisément célébrée ce mardi 17 octobre la France classée parmi les pays dits riches n'échappe cependant malheureusement pas à la pauvreté, puisque près de 9 millions de nos concitoyens souffrent de cette situation, fréquemment, ce sont les mêmes d'ailleurs qui ont à supporter la double peine, être pauvre et stigmatisé trop souvent la méfiance, voire la défiance l'emporte sur la confiance, trop souvent, il est question d'assister, alors que nous devrions parler d'ayant droit de notre démocratie, trop souvent l'isolement et le compagnon de la misère, trop souvent, enfin les complexités administratives sont les causes du non-recours estimée à plus de 10 milliards d'euros par an dans notre France des droits de l'homme, un enfant sur 5 est pauvre et même un sur 2 dans nos zones urbaines sensibles, oui, ceci est condamnable, oui, ceci est intolérable, certes quelques avancées ont eu lieu nécessaire mais toujours très insuffisante face à l'ampleur du fléau c'est d'un véritable plan de lutte pour l'éradication de la pauvreté dans notre société a besoin, c'est cela qu'il faut mettre en oeuvre en liaison étroite avec les associations caritatives et humanitaires et jamais, jamais, la lutte contre la pauvreté ne doit servir de variable d'ajustement budgétaire, quelle est votre ambition sur cette question majeure qui est autant social que sociétal, monsieur le 1er Ministre : quelles mesures comptez-vous prendre mes chers collègues, un illustre prédécesseur au sein de notre assemblée, Victor Hugo écrivait : l'homme est fait non pas pour traîner des chaînes mais pour ouvrir des ailes en s'attaquant sans relâche à ce drame de la misère, c'est tout, si ouvrir un peu plus les ailes de notre démocratie, alors faisons-le.

Voilà un accueil chaleureux, monsieur le président, Monsieur le président, Mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, Vaugrenard, je crois qu'ici dans l'hémicycle, quelle que soit l'endroit où on se situe cet enjeu de lutte permanente contre la pauvreté va tous nous rassembler, parce que le constat et vous l'avez fait et dramatique, 3 millions d'enfants, c'est un enfant sur 5, c'est un enfant sur 5 qui aujourd'hui est dans la situation de grande pauvreté, ces 20 pourcent d'enfants pas de de pauvreté dans les familles monoparentales et si vous êtes confronté à une mère isolée, sans travail, c'est 70 pourcent des des familles qui sont sous le seuil de pauvreté, voilà la réalité, ce que nous connaissons dans notre pays aujourd'hui en ce 17 octobre Mgr ce triste anniversaire, ce 30ème cette 30ème journée internationale de lutte contre la pauvreté et vous a raison : nous devons agir, agir à tous les niveaux, et c'est ce que le gouvernement fait c'est ce que le gouvernement fait en matière d'école quand nous investissons massivement dans les quartiers les plus difficiles de notre République dans les raids plus ou ne des doublons les classes le gouvernement agit aussi en matière de logement et c'est le problème Logement d'abord qui s'adresse à 16 et ceux qui, aujourd'hui, sont exclus du logement sont obligés de séjourner notamment en hôtel pour lequel nous sommes mobilisés le gouvernement agit aussi dans la loi de finances et vous avez raison et vous évoquez l'ISF, je citerais volontiers moi aussi Victor Hugo qui disait : il faut savoir limiter la pauvreté sans limite la richesse celles et ceux qui considèrent qu'on peut dépenser ce que nous n'avons pas produit et ceux qui pensent qu'il faut produire pour pouvoir dépenser pour pouvoir protéger pour pouvoir aider les femmes et les hommes qui sont dans cette grande difficulté et c'est tout le sens de l'action que nous portons dans le projet de loi de finance et je ne doute pas que vous le votiez quand il s'agit de revaloriser revaloriser l'allocation adulte handicapé quand il s'agit de revaloriser les minima sociaux qui n'ont pas été mesdames messieurs depuis 5 ans, c'est ça la réalité du projet de loi de finances, mais le président de la République veut aller plus loin et ce matin il a réuni l'ensemble des acteurs de la lutte contre la grande pauvreté pour définir avec eux et avec ceux qui sont concernés, un plan d'action qui doit tous nous mobiliser. La parole est à notre collègue Daniel Chassain pour le groupe République et Territoires, les indépendants, vous avez la parole monsieur. Président, Monsieur le Ministre, mis, chers collègues, ma question s'adressait à Madame le Ministre des solidarités, de la santé, elle porte sur le sujet, les déserts médicaux : l'absence de médecins condamne des territoires à la désertification, pas de retour de retraités pas d'implantation John pas de touristes, pas d'économie et pas des pharmacies en grande difficulté, les progrès technologiques comme la télémédecine qui constitue un plus pour les médecins ne saurez le remplacer, vous avez proposé, un plan qui va dans le bon sens en pour FIFA incitation maisons de santé avec des actions nouvelles collaborations public-privé Emploi territoire tant médical consultations avancées maître de stage, permettez-moi d'émettre quelques propositions complémentaires augmenter le numerus clausus 20 pourcent des des diplômés ne s'installe, ni remplace et instaurer un internat par faculté en fonction des besoins de du territoire renforcé des stages du 2ème cycle chez le médecin généraliste, instaurer un internat de 6 mois chez le praticien lanterne épaulant le médecin instaurer la mise en place de médecin salarié les souhaite que les jeunes ne souhaite pour intervenir dans les maisons de santé embauché par une association hôpital mairie département ou un j'ai acheté qui évoluerait juridiquement envisager enfin des solutions plus contraignantes non-conventionnement de l'assurance maladie pour les praticiens qui s'installeraient en hyper dense, engagement de l'État pour qu'aucune maison de santé n'aura, sans médecin interne sous la responsabilité d'un médecin référent hospitalier ou intervention d'un jeune diplômé salariés éventuellement sur une période à définir la République doit garantir l'accès aux soins de 1er recours par la présence d'un médecin dans les maisons de santé du territoire, je vous remercie, Monsieur le Ministre, votre réponse, très attendu, notamment dans les zones rurales. Pour vous répondre. La parole est au ministre de la cohésion des territoires que Jacques Mézard. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Daniel Chassain, vous représentez le département de la Corrèze, département béni des présidents de la République et dans lequel il semble qu'il y avait un manque de médecins, je veux ce que je tiens à vous dire parce que je connais bien cette cette problématique cette problématique qui vise non seulement d'ailleurs nombres de territoires ruraux, mais aussi les quartiers fragiles dont nous parlions tout à l'heure, je crois que vos propositions et j'en suis sûr vont dans le bon sens d'ailleurs, je vous prie d'excuser l'absence de Madame la ministre de la santé, mais vous dire que le plan qu'elle a présenté correspond vraiment aux mesures que vous souhaitiez bien sûr nous prendre en considération ce que vous avez proposé, mais le plan correspond à vos demandes, ce plan prévoit prévoit la création de 300 postes d'assistants partagés salariés par l'hôpital qui pourront exercer à la fois dans une structure hospitalière, mais aussi dans des structures ambulatoires dans les zones sous-denses aussi ce qui est prévu, c'est le doublement du nombre des maisons de santé 1000 sur le quinquennat avec 400 millions du plan d'investissement prévu là-dessus aussi des aides à l'installation qui sera renforcée, avec un budget de 200 millions d'euros la possibilité et c'est important dans nos territoires, nous le savons, la possibilité pour les généralistes retraités d'avoir une activité à temps partiel, je crois que ça c'est une bonne chose, un bon signal, vous avez aussi parlé du contrat d'adjoint dans les zones sous-denses qui permet à un étudiant en médecine d'exercer en même temps qu'un autre médecin installé en soutien, ce sont, cet ensemble de mesures auxquelles d'ailleurs peuvent s'ajouter d'autres dispositions qui permettront d'aller dans le sens que vous souhaitez et puis un mot sur le numerus clausus, il faut 10 ans que ça pour que ça produisait fait ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, nous y réfléchissons, mais ça ne résout pas les problèmes à court terme, voilà les quelques éléments que je voulais aller qui vont d'ailleurs dans le sens de votre excellente question Docteur Chassang. Monsieur le ministre avec Madame le ministre de la Santé, soyez les ministres de la République pour la santé ce que Jules Ferry a été pour l'école, en permettant à toutes les maisons de santé d'avoir un médecin pour l'accès de soins de 1er recours dans nos territoires. Merci. Et maintenant, à notre collègue Christophe Priou, pour le groupe, les républicains. Merci monsieur le président. La question s'adresse à monsieur le 1er ministre et concerne le projet d'aéroport du Grand-Ouest de nombreux collègues élus locaux se trouve aujourd'hui confrontés à des citoyens qui, s'inspirant de la note d'implication du droit sur la zone de Notre-Dame-des-Landes règne initiative de s'affranchir si doivent la réglementation, notamment en matière d'urbanisme premières question : comment comptez-vous rétablir l'État de droit, alors même que les élus locaux font face à un phénomène contagieux de désobéissance civile du à l'inertie de l'État 2ème question les médiateurs dits indépendants n'ont pas trouvé le temps d'auditionner collectivités, membre du syndicat mixte de l'aéroport, l'unique contact établi était enfin bref appel téléphonique au maire de Saint-Nazaire à 15 heures pour un un rendez-vous à 17 heures à Nantes, expliquez-nous, Monsieur le ministre, comment a été choisi des médiateurs dits indépendants et en même temps, pouvez-vous nous obtenir le résultat des études complémentaires et comment ont été sélectionnés mandaté les cabinets d'études, le devoir de vérité et de clarté s'impose pour répondre à une population et ces élus qui se sentent floués abusés après un référendum au résultat pourtant incontestable en faveur de la réalisation de cet aéroport. Pour vous répondre, la parole est à madame la ministre. Chargée des transports, Madame Borne. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur Priou je tiens tout d'abord à saluer le travail considérable qui a d'ores et déjà, été réalisées par la mission de mes médiation sur le projet de transfert de l'aéroport de Notre-Dame Atlantique à Notre-Dame-des-Landes, la mission a auditionné plus de 100 50 personnes, selon une méthode qui a permis de nouer le dialogue à la fois avec les partisans du transfert comme avec les opposants et je pense que chacun peut avoir accès à la mission, mais j'ai bien noté les cas particuliers que vous avez évoqué, que je signalerai à la mission, la mission mène un travail d'analyse technique, qui doit mettre en lumière, de manière factuelle impartial les avantages et les inconvénients de chacune des options dans ce cadre, la lettre de mission prévoyait bien quel recours à des expertises qui sont menées sur la base d'un protocole strict et dans le respect des règles de la commande publique ces expertises seront rendues publiques et chacun pourra comparer et analyser les résultats et les méthodes de ces travaux, alors je sais que ces travaux sont suivis avec attention, avec une vigilance toute particulière, tant par les partisans que par les opposants à ce transfert, j'entends les impatiences, mais le moment est à l'analyse et à l'écoute et je pense que chacun, dans un esprit de responsabilité doit permettre à la mission de mener son travail sereinement, je pense que vous pouvez noter que le gouvernement a fait preuve à la fois de diligence et de transparence sur la méthode, dès son arrivée, je rappelle que la mission a été lancée dès le 1er juin soit moins de 15 jours après l'installation du gouvernement son rapport sera remis en décembre prochain pour éclairer les choix du gouvernement sur les options en présence, le gouvernement prendra alors ses responsabilités, je vous remercie. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, vous ne nous avez pas convaincus sur l'indépendance des experts, ils auraient pu être rejoints par d'autres experts aussi indépendant que Madame Duflot Monsieur Mamère GeForce appelle le trait puisque 2 experts sur 3 était notoirement contre le projet actuel avant leur nomination ce ne sont pas les déclarations médiatiques du ministre d'État en charge de la transition écologique et solidaire sur une éventuelle démission mise dans la balance, qui sont de nature à nous rassurer, sinon pour lui-même, à méditer un adage qui avait été prononcée par un ministre, qui fut sénateur également Jean-Pierre Chevènement sur le temps d'ici, c'est la parole ministérielle merci. merci. La parole est maintenant notre collègue. Georges Patient pour le gros de la République en marche. Monsieur le président, chers collègues, ma question s'adresse à la ministre des Outre-Mer. Madame la ministre. Dans une Guyane pas apaisées depuis les derniers événements de mars/avril 2, sujet très brûlant exaspère les Guyanais. Le 1er concerne l'immigration clandestine. Qui se poursuit, qui continue à se poursuit à un rythme effréné, plus de 11000 demandes d'asile recensés dans un pays de 250000 habitants, autant que dans toute la France hexagonale, à telle point que certains dans le pays, n'hésite pas à parler de génocide par substitution, le second sujet de crispation porte sur le respect des accords de Guyane avec leur absence de visibilité dans les documents budgétaires et dans le grand plan d'investissement je veux espérer que le président de la République, qui se rend en Guyane, en fin de semaine prochaine apportera à la population guyanaise, les réponses attendues ce sont sur ces 2 questions incontournables, mais aujourd'hui je voudrais surtout traiter du dernier rapport de la Cour des comptes, d'une violence inédite à l'égard des élus d'outre-mer. Dans la foulée de cette charge, le président de la chambre régionale des Antilles Guyane sortant de son rôle car se sentant la population à sanctionner les élus. En outre, mer, tout paraît permis une telle posture de la Cour des comptes est d'autant plus désolante que ce rapport est parsemé d'erreurs grossières. En effet, pour étayer sa démonstration, qui consiste à dire que les collectivités d'outre-mer sont très riches, mais que leurs difficultés financières découleraient uniquement d'une mauvaise gestion, la cour n'hésite pas à faire des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être, pourquoi donc une telle charge alors que l'on sait que les collectifs d'outre-mer sont au contraire dans une impasse budgétaire structurel pour masquer les graves manquements que subissent les communes d'outre-mer, au niveau de la péréquation. La cour finit tout de même par le reconnaît dans son rapport pour la première fois, alors que depuis 10 ans, les villes capitales des Outre-mer et moi-même ne cessons de le clamer haut et fort : il s'agit cependant d'une avancée majeure, votre question. les 2 questions sont les suivantes. Alors quel train de vie peuvent mener des communes de des Dom dans un contexte de pénurie financière. Et madame la ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour que, dès 2018 les communes des domaines bénéficient d'une péréquation juste et équitable. Merci madame la ministre avait 2 minutes. minutes. Il appelle. Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, la Cour des comptes, vous l'avez dit, a mis en lumière dans son dernier rapport, une situation financière des collectivités locales plus dégradée dans les départements d'outre-mer quand métropole en cela, elle est dans son rôle et je ne ferai pas de commentaire sur ces conclusions par compte je veux comme vous affirmer ici que les collectivités d'outre-mer sont confrontés à des défis propres que le débat sur leur situation financière ne peut absolument pas, et vous avez raison d'en parler, c'est vrai pour la Guyane où l'explosion démographique ou la taille encore des communes constituent des enjeux majeurs pour lesquels les collectivités sont insuffisants, mon armée et je le rappelle à tous des collectivités qui sont seuls à connaître ce type de défi aujourd'hui en France, les accords de Guyane en avait parlé en d'ailleurs traduit l'engagement et la solidarité du gouvernement en 2017 avec 89 millions d'euros supplémentaires qui ont été fléchés pour la collectivité territoriale et pour les communes qui bénéficieront pour leur part d'un surcroît de recettes liées à l'octroi de mer qui s'élèvera à terme à 27 millions d'euros, plus généralement, l'ensemble des territoires d'outre-mer vive au quotidien l'éloignement, l'insularité ou l'enclave en et connaissent des taux moyens de pauvreté et de chômage sans équivalent dans l'Hexagone et là aussi je vous rejoins dans ce cadre, la conférence nationale des territoires que le gouvernement a lancé mène une mission chargée de proposer un contrat de mandature aux collectivités et je veille à ce que les particularités de l'mer soient bien prises en compte et j'ai moi- même pour alimenter par des données bien spécifique, ces débats, demandé à ce qu'un travail soit fait sur les structures décharger des recettes des collectivités ultramarines et ce rapport sera nous sera rendu au 1er semestre 1018 et nous pourrons en partager les chiffres de manière à ce que les choses soient claires et bien comprise, monsieur le sénateur, je le dis souvent : je n'ai pas de sujet tabou et ma méthode et la transparence et nous continuerons effectivement à la mener, l'enjeu est clairement posé les termes du débat doivent être équilibrées, les chiffres précis et nous aurons tous ces débats. Merci, la parole est à notre collègue Pierre Cuypers pour le groupe, les républicains. Monsieur le président, ma question s'adresse à monsieur le 1er ministre monsieur le 1er ministre la MSA dénonce qu'en 2016 un tiers des agriculteurs français a gagné moins de 350 euros par mois, l'urgence est donc déclarée dans le contexte actuel des états généraux de l'alimentation, le président de la République a formulé un certain nombre de propositions et je cite : redonner du pouvoir d'achat nos agriculteurs en leur donnant la possibilité de proposer eux-mêmes un contrat au groupe agroalimentaire avec une prise en compte des prix de production et avec la mention obligatoire des coûts de revient dans les contrats de soutenir également en outre le relèvement du seuil de revente à perte ces dispositions seront possibles, selon lui, si les agriculteurs se structure en filière et on forte portant chacune un projet de transformation, permettez-nous d'en douter, pour le moment, la nature et le calendrier de ces engagements sont très approximatifs et reste bien évidemment à définir, changer les modèles productifs peut-être mais un arrêt comme il a été dit par le président de la République de certaines productions ne s'inscrivant pas dans la concurrence internationale serait catastrophique et fatale attention de donner à l'agriculture, les moyens de cette compétitivité monsieur le 1er Ministre merci de préciser comment le gouvernement entend donner suite à ces propositions, faire état d'un calendrier renvoyer les modes d'application prochaines années serait un mauvais signal. j'ai bien entendu votre question est certainement comme moi, vous avez été attentif au discours du président de de la République, un discours qui redonne du souffle à notre agriculture, un discours qui veut faire en sorte que les agriculteurs demain puissent vivre dignement de leur revenu et pour que les agriculteurs puissent vivre dignement de leur revenu, nous nous appuyons sur plusieurs volets : d'abord la construction du prix oui, il faut revenir à une inversion du prix en faisant en sorte que l'on parte du prix de revient des producteurs pour mécaniquement remonter ensuite chez les transformateurs et les distributeurs afin que chacun puisse être rémunérées à la juste valeur ensuite le président de la République a prononcé et a souhaité que les agriculteurs puissent se regrouper en organisations de producteurs pour avoir plus de force pour que le triptyque, transformateurs, distributeurs, producteurs puissent être un triptyque gagnant gagnant gagnant et, enfin, d'ici la fin de l'année, nous présenterons au président de la République avec le travail des filières, un plan de filières, un plan de restructuration des filières qui devra nous permettre demain d'avoir des filières mieux armé pour répondre à la concurrence européenne et mondiale, avoir des filières qui puisse avoir une vision d'avenir des filières qui peuvent investir des filières qui peuvent innover, c'est cela le visage de l'agriculture de demain, c'est cela le visage de la ferme France que nous souhaitons demain pour notre pays et nous avons ainsi bouclé quelque part le chantier numéro un sur la création et la répartition de la valeur et nous souhaitons, Monsieur le Sénateur, vous le savez bien, à travers le 2ème chantier que nous allons d'ores d'ores et déjà mis en chantier en oeuvre ces derniers jours, hé bien faire en sorte que nos consommateurs puissent avoir une alimentation saine, durable et accessible à tous, c'est miser sur la qualité, c'est monté en premium, la gamme 2 aux aliments en faisant en sorte que le budget moyen du consommateur ne soit pas altéré et pour cela, nous disposons d'un certain nombre d'outils, il faut commencer dès le 1er semestre prochain, nous nous engageons à travers un projet de loi pour faire en sorte que la ferme France demain soir au rendez-vous de ces défis et des enjeux qui l'attendent, merci monsieur.

et d'avoir les politiques qui les accompagnent, qui les soutiennent et non qui les entravent merci. La parole est à notre collègue Angèle Préville pour le groupe socialiste et républicain, vous avez la parole. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, cette question, ça s'adresse à Madame Schiappa longtemps les femmes se sont tus parce que le moyen de survie en milieu hostile, et d'être comme étranger à soi-même les femmes en face de dissociation après une agression, ne parlent pas la parole des femmes c'est libéré donc face à la clameur obtenues par résonance des dizaines de milliers de truites, que comptez-vous faire, Madame la Ministre, ce cri qui s'étouffer dans nos gorges, le voilà enfin audible par le truchement des réseaux des il est considérable, il doit être non seulement entendu, mais pris en compte vraiment accompagnée de mesures concrètes, rapides au secours des femmes qui ont osé s'exprimer mais agir ne doit pas être seulement panser les plaies, il faut s'attaquer aux racines du mal, peut-on envisager un débat de moralisation générale qui permettrait de questionner la pornographie accessible à tous et notamment à nos enfants la publicité qui entretient l'idée que nous les femmes sommes des objets d'envisager un volet pédagogique d'information aux filles absolument nécessaire est cruellement absent sur les dangers à être une fille, une femme dans notre société, sans oublier l'éducation des garçons qui doit être conjointe qu'allez-vous envisagez concernant ces hommes de pouvoir ayant abusé de leur position dominante pour contraindre les femmes à ce qu'elle ne voulait pas, je me prends à rêver, c'est un rêve subversif que les entreprises, les administrations pour les dans lesquelles des présidents des directeurs des chefs d'équipe ont fauté, voient leur poste forcément remplacés par une femme et, enfin, je pense aux femmes qui ne peuvent s'exprimer, je veux parler des femmes qui sont victimes de violences qu'on dit pudiquement conjugale, c'est un Crime de masse qui est passé sous silence et qui concerne environ 130 femmes par an, que proposez vous de concret pour diminuer le nombre de ses victimes peut-on envisager ce qui serait une déjà une solution une médiatisation, à la fois national, c'est-à-dire une information claire dans les journaux

à la secrétaire d'État, Serge et de l'égalité entre l'homme et les femmes Madame Marlène Schiappa avait lapin. Merci Monsieur le Président, Madame la sénatrice, mesdames et sénatrice, messieurs les sénateurs, vous avez extrêmement bien posé la question à madame la sénatrice, je vous remercie pour votre engagement, que pouvons-nous faire c'est une vraie question parce que, encore, les femmes parlent, ça ne suffit pas qu'elle parle, encore faut-il que la société les entendez que les pouvoirs publics leur répondent c'est pour leur répondre que le président de la République a décidé que l'égalité entre les femmes et les hommes étaient la grande cause nationale de son quinquennat c'est pour répondre aux femmes que nous augmentons le budget des droits des femmes pour 2018 et ou, sans nous le sanctuarisant pour l'ensemble du quinquennat et c'est pour répondre aux femmes que le 1er ministre a lancé le 4 octobre dernier le Tour de France, de l'égalité entre les femmes et les hommes, les ateliers, les consultations de ce Tour de France nous amèneront à déposer en 2018, un projet de loi une première grande loi citoyenne à cet égard que je présenterai avec la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, cette loi qui associera tout le monde, les parlementaires, les territoires, les experts, les victimes, les femmes, les associations nous permettra de répondre et d'assurer une juste condamnation sociétal et judiciaire des violences sexistes et sexuelles pour terminer si je partage pleinement, Madame la sénatrice, votre engagement sur le fond je me permettre une petite réserve sur la forme, je ne pense pas qu'il s'agisse de morale, je pense qu'il s'agit d'autres droits Nietzsche disait il n'y a pas de phénomène moraux, il n'y a qu'une interprétation morale des phénomènes, je pense qu'il s'agit de droit et que c'est pour cela que nous devons faire évoluer notre droit et que je compte sur les sénatrices et les sénateurs pour cela je vous remercie. Je Je voudrais remercier le 1er ministre ensemble des ministres, je vous rappelle que les prochaines questions d'actualité au gouvernement auront lieu le 26 octobre seront retransmis sur France 3 Public-Sénat et notre site internet, je vais suspende la séance, elle sera reprise à 17 heures 50 pour la la suite de notre ordre du jour séance est suspendue.

Chers collègues, la séance est reprise. Nous reprenons la discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance du Diffé vrier 2016 portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations dans la discussion des articles, nous sommes parvenus à l'article 6. Nous sommes à l'amendement numéro 28 qui n'est pas soutenu, je ne vois pas, mais ceux

Bien alors monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le rapporteur, donc sur ce point-là, c'est-à-dire sur la nécessité de préciser la définition de la capacité des personnes morales, nous partageons la position de la Commission. Le gouvernement n'avait aucunement souhaité en consacrant la capacité des personnes morales dans le code civil modifié le droit positif, la référence aux actes utiles à la réalisation de l'objet statutaire ne visait nullement à exiger une appréciation en opportunité de l'acte au regard de l'intérêt social de la même manière, le gouvernement n'entendait pas par ce texte, remettre en cause les solutions propres à chaque forme de personne morale, j'ai entendu toutefois les craintes qui ont été émises par les praticiens sur la porte et qui pourraient être données à ce texte une réécriture du texte pour poser le principe de capacité limitée des personnes morales et renvoyer au texte, propre à chaque personne morale me semble donc je vous propose toutefois un amendement de nature purement rédactionnel, afin de préciser le renvoi opéré aux règles spéciales pour qu'il soit prévu, je cite, que la capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles. Merci madame la garde des Sceaux, avis de la commission. après un échange avec les services de la chancellerie, je dois avouer, dans ces conditions, que ne comprend pas bien pourquoi cette rédaction ne convient pas ou ne convient plus, d'autant que la rédaction proposée par le gouvernement, par un peu restrictives, dire que la capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'elles supposent qu'il existe bien des règles claires, écrites, qui n'est pas évident, droit des sociétés, contrairement aux droits des associations, la formulation retenue par la commission ne sont plus large, plus adaptée à cette diversité des droits spéciaux en mentionnant dans le respect des règles applicables à chacune d'entre eux. Je dis donc, j'ai trouvé le le le travail de la commission, peut-être un peu plus ciselée, pour autant, il ne paraît, il ne m'apparaît pas compte tenu de des termes de votre rédaction et du fait que vous avez effectivement noté ces difficultés que votre amendement soit de nature. à mettre une écharde entrent dans nos relations, c'est la raison pour laquelle j'ai être un avis de sagesse, je viens de sagesse positive.

qui est pour. L'article 6 être adopté, nous passons à l'article 7. Avec 3 amendements, ce sont l'objet d'une discussion commune. L'amendement numéro 10 Madame Mellow. Si Monsieur le Président, le nouvel art. Cycle 1128 du code civil, supprime la référence à l'accord et à l'objet du contrat remplacé par la notion de contenu du contrat, les nouveaux articles 1162 à 1171 du code civil décline cette nous Sion reprenant ont une partie des différentes fonctions que la jurisprudence avait assigné à la cause et à l'objet. Il s'agit de concept précis, défini par une abondante jurisprudence mais également de notions suffisamment ce flexible pour permettre au juge de s'adapter à l'apparition de nouveaux risques contractuels et de nouvelles situations, or l'ordonnance remplace concepts tout à la fois précis et souple par une notion floue et incertaine, celle de contenu du contrat qui ne marquera pas, qui ne manquera il convient de souligner que la suppression de la cause a été juste, justifiée par le faux prétexte que celle-ci aurait nui à l'attractivité du droit français, or aucune entreprise étrangère ni aucune entreprise étrangère dans ses rapports avec des partenaires étrangers n'a jamais refusé l'application du droit français, afin d'échapper à la cause, il convient dès lors de rétablir les notions d'objets et de cause à la place de celle de contenu, le nouvel article 1162 du code civil doit également être modifié pour faire référence à l'objet et à la cause du contrat.

oui Monsieur le Président, c'est un moment de 2 séances comme les autres, à l'exception du 30, les autres ont été discutés en commission ce matin et sont tous retirés à l'exception du 30. Je comprendre tout à l'heure. L'avis

la cause du contrat en particulier toutes les générations d'étudiants en droit, dont je suis, bien qu'elle serait peut-être assez prête à confesser que même au bout de 10 ans Les et contours de cette théorie ne lui sont pas totalement acquis, les représentants de certains systèmes juridiques étrangers très inspiré par notre code civil c'est particulier, ceux de l'armée grecque, latine ou de l'ou du Liban, nous en font également le reproche toutefois la doctrine a majoritairement, me semble-t-il valider cette évolution que certains appelleront une modernisation, surtout si la cause a disparu, il me semble que les éléments constitutifs sont toujours présents, d'une part, l'article 1128 précise que le contrat doit avoir le un contenu licite et certains pour être valide, et l'article 1162 indique qu'il ne peut être il ne peut pas l'déroger être dérogé à l'ordre public par son but, le contenu et les but renvoie en fonction de la cause, de sorte que la jurisprudence ne doit pas s'en trouver bouleversée jeudi en commission ce matin pour prendre une image, peut-être un peu légère que la cause était sortie côté jardin était rentré, côté cour et que peut-être ça ne méritait pas que l'on modifie sur ce point l'ordonnance je rappelle d'ailleurs la ligne générale de la commission, le Sénat était hostile à une aussi importante réforme de notre droit civil par ordonnance, mais maintenant que la réforme est en vigueur depuis plus d'un an, nous devons faire preuve de responsabilité et de ne pas remettre en cause les grandes solutions de la réforme et la suppression de la cause en est une, sinon les praticiens ne comprendraient pas, j'espère, si je ne vous ai pas convaincu de vous avoir rassurés sur le fait que, dans l'ombre la cause existe encore et que de ce fait, vous pourriez peut-être votre amendement. Merci, monsieur le rapporteur.

donc tant qu'il n'a pas vocation à s'appliquer dans les champs déjà couverts par des dispositifs comparables en droit de la consommation est en droit de les relations commerciales, le géant du droit allemand peut légitimement nourrir vos critiques, on peut aussi critique This critiqué dispositif car le droit commun des contrats postule l'égalité entre les partis et les déséquilibres structurels sont traitées par les droits spéciaux par esprit de responsabilité auquel je vous invite vous associer la commission n'a pas remis en cause ce choix du gouvernement qui semble admis. Certes, sans grand enthousiasme et admis par les milieux économiques dans le périmètre qui est circonscrit, des contrats d'adhésions dont la commission a revu la définition à l'article 1100 et là aussi, je vous suggère de retirer cet amendement sans pour autant renoncer ou la motivation assez réelle et sérieuse que vous aviez proposé. Merci, monsieur le rapporteur de l'avis du gouvernement dans la galerie, sur les 2 3 et ma vue Maranello Messier donc accepter de retirer vos amendements. Je voudrais remercier monsieur le rapporteur, pour toutes les précisions qu'il a apporté, bon je ne suis pas membre de la commission des lois, donc je n'avais pas entendu tous tous ces arguments, je vais retirer et les amendements merci.

ambiguïté en toute ambiguïté relatives à l'identité du co-contractants qui peut se voir octroyer une prérogative de fixation unilatérale du prix, il convient de préciser que dans les contrats cadres il y peut-être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par le fournisseur de bien ou. Le prestataire de services,

le débiteur de l'obligation qui puisse fixer unilatéralement le prix, l'inverse est sans doute un cas d'école, une hypothèse assez rare, cet amendement donne l'occasion de clarifier cette interprétation sans modifier le texte, en outre, l'article 1164 précise que les parties peuvent en disposer ainsi, c'est-à-dire qu'elles peuvent aussi ont disposé autrement : c'est une disposition supplétifs de volonté, donc on peut y parer par une disposition sur ce point, en d'autres termes, laissons les partis décider librement qui peut fixer le prix dans un contrat cadre, que ce soit le débiteur ou exceptionnellement le créancier, je pense que ça peut ne pas vous inquiéter et là encore je vais solliciter un retrait.

à l'amendement numéro 5 rectifier bis toujours Madame Mellow. Je vais, je persiste et signe, donc là il s'agit de d'insérer un alinéa ainsi rédigé à la première phrase le mot créanciers et remplacé par les mots prestataires de service.

H 56 de mon rapport, c'est un amendement donne l'occasion de clarifier l'interprétation qui est affaire de cette disposition, dont acte, et dès lors, il n'y a pas à modifier le texte donc demande de retrait.

Ce texte permet de fixer le degré de qualité de la prestation attendue dans un contrat lorsqu'aucune clause ne la détermine ni ne permet de la déterminer l'ordonnance s'inspire d'ailleurs sur ce point des projets européens d'harmonisation du droit qui renvoie aux attentes légitimes des partis, c'est-à-dire de toutes les parties au contrat. En effet, la qualité de la prestation doit être appréciée tente au regard de ce que le créancier pouvait espérer recevoir mais également de ce que le débiteur s'attendait de son côté à devoir fournir la présentation qui a été faite par le rapport au président de la République était destiné à illustrer l'intérêt de ce texte, elle ne doit donc pas être interprétée comme limitative lorsqu'elle ne renvoie qu'à la qualité attendue par le créancier, les sommes attendues créanciers ne constitue pas le seul élément d'appréciation de la qualité de la prestation qui doit être effectivement recherchées dans la commune intention des partis au regard du type de contrat en cause selon les circonstances de sa conclusion à une mise en une mise en balance des attentes respective des partis qu'invite à procédé le texte d'ailleurs en visant, je cite, les attentes légitimes des partis, l'article 1166 entendait se démarquer de l'ancienne Artic. 1246 du code civil qui ne renvoyé lui qu'à la seule situation du débiteur, en outre, le recours à la notion d'attente légitime des parties permet d'objectiver l'appréciation de la qualité de la prestation en l'absence de stipulation contractuelle sur ce point, le contenu de cette notion d'attente légitime sera notamment déterminer en considération de la nature de la prestation cause des usages dans le domaine et de la contrepartie, c'est-à-dire le plus souvent du prix. Il nous sommes préférable, donc dans un souci d'équilibre, de ne pas s'attacher aux seuls attendu créanciers, c'est donc au bénéfice de ces explications que je vous demanderai de bien vouloir rétablir le texte initial de leur. Oui, Monsieur le Président, j'ai un peu de mal à suivent le raisonnement du gouvernement sur la rédaction initiale de l'ordonnance sur ce point, pourquoi, pourquoi il veut y revenir l'ordonnance indique lorsque la qualité de la prestation n'est pas déterminée ou déterminé à blanc, fonction du contrat que le débiteur de l'obligation doit fournir une prestation de qualité conformes aux attentes légitimes des pas, je ne comprends pas, quelle peut-être l'attente légitime pour le débiteur de l'obligation, en terme de qualité de prestations, il est le mieux à même de savoir ce qu'il peut attendre de lui même, c'est bien le créancier de l'obligation qui peut légitimement, attendent un certain niveau de qualité incertitude type de prestations tempéré d'ailleurs par la nature de la prestation, les usages de la profession et le prix 3 critères indiqués par le code civil qui constituent autant de critères d'objectivation qui guideront le juge si besoin, devant la commission des lois, j'ai pris un exemple qui comme toute exemple peut-être certainement contourner et amener de contre exemple lorsque vous commandez votre portrait, un, il peut être plus ou moins ressemblants voire plus ou moins figuratif et il est difficile de déterminer précisément la prestation dans le contrat, l'attente légitime celle de celui qui commande le portrait. Pas celle du peintres, alors je ne comprends pas donc pas la signification de la référence aux attentes légitimes des 2 parties sur ma proposition de la Commission avait retenu une rédaction qui m'apparaissait plus clair sans utiliser la notion inusité d'attente légitime et en se calant d'ailleurs au plus près de l'objectif énoncé sans ambiguïté dans le rapport au président de la république qui dit que la qualité de la prestation qui ne peut être déterminée à l'avance doit correspondre, c'est le rap dans le rapport au président de la République lui-même le dit, à la qualité que le créancier pouvait raisonnablement espérer c'est la région. Pour laquelle je félicite Madame la Garde des Sceaux, le retrait de votre amendement et puisque je ne recèle j'ai, à défaut, un avis défavorable.

Oui, merci Monsieur le Président, il s'agit là d'un d'un amendement qui, s'il était peut-être adopter bouleverserait l'économie générale du texte, d'une manière assez relative puisque il s'agit tout simplement de supprimer quelques mots la seconde phrase de l'année est à un an de l'article 1183 la cause de la nullité doit avoir cessé tout simplement parce que s'il s'agit d'une nullité subjective, évidemment, elle doit avoir cessé sinon elle hier et la confirmation qui fait l'objet de de l'article, il s'agit du vice de consentement, tels que l'erreur le Dol ou la violence, évidemment, elle doit avoir cessé à défaut

et on pratique le texte et au regard de la de la jurisprudence finalement interdit de de confirmer l'acte et donc ces quelques mots sont devenus superfétatoire et cet amendement tout simplement propose de lier voté hôtels du texte.

puis après réflexion, j'ai renoncé à modifier le texte, le code prévoit ce qu'on appelle une action interpellative dans l'hypothèse où un contrat est entaché d'une cause de nullité une partie peut demander à celles qui pourraient se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat, soit d'agir en nullité dans un délai de 6 mois, ce dispositif a pour but de purger le débat sur la nullité notre droit ne cesse de trouver des techniques pour purger les nullités pour sécuriser le contrat ou bien éventuellement, pour demander l'annulation, pourquoi est-il logique de prévoir que la cause de nullité doit avoir cessé pour que cette action interpellative puissent être mises en oeuvre, je précise que ceci vaut pour les cas de nullité relative car on ne peut pas confirmer un contrat entaché d'une nullité absolue, l'objectif est de protéger la partie qui pourrait se prévaloir de la nullité pour faire annuler le contrat pour éviter qu'elle ne soit atteinte par la forclusion de l'action en nullité, tout ça est très technique, dans les 6 mois d'interpellation si l'autre partie à l'origine de la nullité l'interroge, par exemple en cas de vice du consentement du fait de violences ou du fait d'un Dol, qui demeure cachée si le con contractant le contractant pardon peut interroger le co-contractants toujours soumis à une situation de violence ou toujours ignorant du dont il est victime, c'est-à-dire une hypothèse dans laquelle la nullité n'a pas cessé, celui-ci pourrait être contraint de confirmer le contrat sans plus être en mesure de se prévaloir de sa nullité ultérieurement, voilà ce qui fait les raisons pour lesquelles, après avoir beaucoup réfléchi par votre question est pertinente, j'ai renoncé à modifier ce texte et j'en reste là, avec l'accord de la Commission, c'est donc comme je vous l'ai indiqué ce matin sur une demande de retrait soit un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur, l'avis du gouvernement, Madame la Garde des Sceaux. je, pour une fois, monsieur le président, je ne partage pas l'avis de monsieur le rapporteur, je rejoindrai assez volontiers la proposition du sénateur de né. L'article 1183 permet à une partie qui a connaissance d'une cause de nullité affectant le contrat et dont pourrait s'par prévaloir un jour ou l'autre partie de lui demander de prendre position afin de régler, sans attendre le sort du contrat, ce texte permet de sécuriser la transaction, l'autre partie disposera en effet d'un délai de 6 mois, soit pour confirmer le contrat, c'est-à-dire renoncer à l'action en nullité soit pour agir en nullité l'exigence selon laquelle la cause de nullité doit avoir cessé visait à empêcher que le co-contractants quelconque tractant pardon, toujours sous l'emprise de la violence, ou qui n'auraient pas connaissance de son erreur, puis se voir imposer la confirmation du contrat, comme le relève, Monsieur le Sénateur de Belenet cette condition peut-être toutefois mal comprise, pour certaines causes de nullité par exemple le non-respect d'un formalisme protecteurs ou le caractère dérisoire de la prestation de l'autre partie, elle doit en réalité être lus à la lumière de l'article 1180 2 qui définit ce qu'est la confirmation, celle-ci n'est admise que si celui qui pourrait se prévaloir de la nullité agi en connaissance de la. Causes de nullité et en cas de violence si celle-ci a cessé, il va de soi que le texte n'exige pas que le contrat soit régularisée, mais seulement que le contractant que la loi vise à protéger et tu pleinement connaissance de la cause de nullité affectant le contrat l'amendement déposé par Monsieur le sénateur de belles n'est en vente, a supprimé cette condition permettrait de lever toute ambiguïté sur la portée du texte, en application de l'article 1182 la confirmation des de toutes façons possibles que si la clause de la cause de nullité est connu et en cas de violence si celle-ci a cessé, je vous invite donc à adopter cet amendement. Merci madame la garde des Sceaux, je vais à présent mettre aux voix l'amendement train très bis qui fait l'objet d'un avis défavorable de la commission est d'un avis favorable du gouvernement il y a-t-il des explications de vote. Il y a maintenant. Pour cet amendement. amendement. L'amendement 30 rectifier n'est pas adopté. Nous passons à présent à l'article 8. Mais cette belle mais j'ai cru comprendre que vous avez retiré l'amendement 31 merci, nous passons à l'amendement 12 rectifier bis, défendu par Madame mélo. Merci monsieur le président, le nouvel article 11 4 11 195 du Code civil introduite en droit positif, la théorie de l'imprévision qui permet de réviser les conditions convenues en particulier le prix en cas de changement de circonstances imprévisibles, la proposition de la commission des lois de supprimer le pouvoir de révision du juge en cas de prévisions va dans le bon sens, cependant, la commission des lois n'a pas proposé de modifier les conditions de l'imprévision pour les encadrer davantage, or la consécration de la théorie de la prévision a pour effet d'affaiblir la portée de l'accord des parties et la sécurité juridique qui est, qui est attachée l'utilité pratique cette disposition apparaît discutable dans la mesure où les contrats entre professionnels prévoient quasiment systématiquement que l'une des parties assument le risque d'un changement de circonstances imprévisibles et où les contrats de consommation sont assorties d'un droit de résiliation unilatérale d'ordre public en faveur du consommateur, il conviendrait dès lors d'encadrer strictement la mise à 9 heures la mise à 9 jours de la théorie de l'imprévision. Merci Madame Mellow l'avis de la commission. Illicitement, voire même expressément à rétablir la notion de cause sur laquelle nous sommes exprimés tout à l'heure, je demanderai donc les mêmes causes produisant les mêmes effets de vouloir procéder bien vouloir procéder au retrait de votre amendement après vous avoir remercié sur l'intérêt des dès qu'il y a à débattre avec vous, puisque vous avez à plusieurs reprises, admis de retirer votre amendement ce qui aussi est un signe, quelquefois, même souvent de responsabilité, j'ai ajoute mais remerciements pour avoir dans votre amendement traduit le droit allemand. Merci messieurs rapporteur même avis pour le gouvernement. Oui, mais ma vie, monsieur le président. Merci madame la garde des sceaux Madame Mellow. Je retire l'amendement je remercie Monsieur rapporte. Merci, cher collègue, nous passons actuellement à 2 amendements identiques le de rectifier bis. Défendu par monsieur Colombain chers collègues.

de cette révision, c'est de rétablir ou d'établir une équité de, de, de, de situation entre les contractants, en l'espèce, qu'est-ce qui est à l'origine de cette, de ce déséquilibre, est sur ce sont. Est survenu pour des des raisons que tout à fait imprévisible des événements extérieurs qui change les conditions dans lesquelles le contrat est conclu, donc nous souhaitons en rester à la rédaction antérieure, celle de l'ordonnance l'idée selon laquelle il s'agirait d'Essat reviendrait à faire intervenir un 3ème parti partenaire au contrat 3ème acteur, qui est le juge

les contrats qui était conclu dans le dans le cas du compte du du code monétaire et financier, initialement, je m'en étais ému, je vois pas pourquoi les exclure, mais à la réflexion, le rapporteur a raison : il s'agit là de contrat tout à fait particulier dans la mesure où effectivement les spéculateurs jouent sur l'imprévisibilité pour retenir un certain bénéfice voilà donc l'idée générale, donc c'est de rétablir la de rétablir le l'esprit

Oui, monsieur le président merci, monsieur rapportant Monsieur sénateurs, que l'on va, mesdames et messieurs les sénateurs, l'amendement proposé par le gouvernement vise effectivement à rétablir la rédaction initiale de l'article 1195 issu de l'ordonnance la rédaction de l'article 1180 15 introduit comme vous n'avez expliqué Monsieur sénateur. La révision pour imprévision dans le droit français des contrats et c'est l'une des dispositions sans doute les plus emblématiques de cette ordonnance du 10 février la France était en effet l'un des derniers pays à ne pas accueillir en Europe, la théorie de la prévision qui était déjà accueilli par le juge administratif d'ailleurs l'objectif de cette innovation et de permettre le rétablissement de l'économie générale du contrat telle que voulue par les partis partis qui aurait été bouleversé, en cours d'exécution du contrat par des circonstances exceptionnelles, il n'est en effet pas équitable au nom de la force obligatoire du contrat et en raison d'un changement de circonstances indépendantes de leur volonté et qu'elle n'avait donc pas prévu de maintenir les partis dans une situation contractuelle déséquilibrées par rapport à leur volonté, exprimée lors de la conclusion du contrat, la possibilité de révision du contrat en cas d'imprévision est toutefois très encadrée et elle ne constitue qu'une dérogation exceptionnelle au principe de l'intangibilité du contrat, tout d'abord le changement de circonstances doit être imprévisible lors de la conclusion du contrat ensuite l'exécution du contrat doit devenir. Excessivement onéreuse pour la partie, ce qui exclut l'hypothèse du seul surcoût enfin à la partie lésée par le déséquilibre ne doit pas avoir acceptées contractuellement d'assumer le risque d'untel, changement de circonstances des inquiétudes nées en raison du pouvoir ainsi conféré au juge, saisi par une seule partie ont sans doute motivé l'amendement de la commission sur lequel je vous demande, mesdames et messieurs les sénateurs de revenir, il faut en effet relativiser l'atteinte portée à la force obligatoire du contrat et à la liberté contractuelle, d'une part. L'article 1195 et supplétifs de volonté, c'est-à-dire que les partis sont libres d'en écarter l'application totalement ou partiellement et de prévoir qu'elles assumeront tous ou certains changements de circonstances modifiant l'équilibre du contrat, d'autre part, les pouvoirs du juge sont strictement encadrées par les principes de procédure civile, le juge ne pourra, d'office, procéder à la révision donc du contrat et il sera, au surplus, lié par les demandes des parties quant à l'objet de la demande et aux modalités de révision du contrat, enfin, conditionner la révision du contrat par le juge à une demande en ce sens, de toutes les parties au contrat réduirait considérablement l'effectivité du textile est en effet très peu probable que des partis qui ne se sont pas entendus sur les termes de la renégociation de leur contrat, voire sur la nécessité. Et même de le renégocier, s'accorde finalement pour en confier la révision au juge, seule la résolution judiciaire du contrat serait alors possible, tandis que sa révision aurait pourtant permis sa survie, ce qui bien entendu présenterait assurément bien plus d'intérêt économique, d'ailleurs, le pouvoir de révision judiciaire accentue l'aspect préventif du texte, le risque de révision du contrat, en plus de celui de son anéantissement devant inciter les parties à renégocier et donc à maintenir le contrat, je vous demande donc de revenir à la rédaction initiale de l'article 1195 et de restaurer la possibilité pour une seule partie au contrat d'en solliciter la révision par le juge. En revanche, le gouvernement ne s'opposera pas à l'exclusion, proposé par le la Commission au grand 2 de l'article 8 de l'application de l'imprévision au contrat sur instruments financiers en effet des risques induits par une telle option paraissent plus fort que les gains espérés, les opérations sur titres financiers sur contrats financiers ont par nature pour objectif d'intégrer le risque dans leur valorisation et dans les caractéristiques retenues pour l'opération, c'est pourquoi je le redis : le gouvernement n'est pas opposé à la rédaction adoptée par la commission sur ce point dans le triple objectif de clarifier clarifier l'application de l'imprévision aux instruments financiers en excluant explicitement les titres et les contrats financiers, sécuriser les transactions futures sur ces contrats, et dernier point contribué par ces 2 actions à l'attractivité juridique de la place de Paris. Merci madame la garde des sceaux qui est l'avis de la commission. Non, premièrement, une question, j'ai à répondre à 2 amendements Certif sont identiques, mais ce que je peux considérer que j'ai 4 minutes. Merci beaucoup 1er point est un point d'ordre si j'ose dire je, je salue la lucidité de notre collègue Colomba lorsqu'il estime que quelquefois le rapporteur peut avoir raison

important, il me semble que le gouvernement a excédé le Champ de l'habilitation législative consentis par le Parlement sur ce point, puisque la loi d'habilitation prévoyait la possibilité pour les partis et non pour une seule d'entre elles, d'adapter le contrat en cas de changement imprévisibles de circonstance. 1er point 2ème point le rôle du juge, c'est bien plus essentiel. J'ai suggéré à la commission qui m'a suivi sur ce point, de ne pas adopter le rôle du juge-t-elle qu'il est prévu dans l'ordonnance, en présence d'une modification radicale du rôle du juge dans nos institutions judiciaires, le juge est son travail c'est d'interpréter un contrat au regard des lois existantes, des règles existantes droit public ou autres et d'analyser comment il doit être exécuté c'est de trancher un litige qui souvent est né dans le passé. Le travail du juge, ce n'est pas de refaire le contrat parce que dans ce cas-là qu'est-ce que devient le juge qui devient économiste, il devint sociologue et au besoin devient fiscaliste et là, l'Euro, le juge rentrent dans une activité qui n'est pas la sienne, et je vais prendre un exemple avec le droit administratif pour faire sentir ce que pourrait être la responsabilité du juge en matière d'acte anormal de gestion très souvent devant les tribunaux administratifs et même pendant très longtemps sous la critique ou la proposition de différents commissaire au gouvernement, dont un à Vernon extraordinaire puisqu'il s'appelait racines, il a toujours été indiqué que les juges administratifs devaient faire très attention pour décider qu'il y avait un acte anormal de gestion, parce que, ce faisant, il. Dans Dans l'exploitation de l'entreprise dans les décisions de l'entreprise et qui prenait une responsabilité qui n'est pas la sienne aussi, moi je vous dis que moi personnellement je pense qu'il ne faut pas intégré dans notre droit, ce rôle très nouveau pour le juge 2ème point Ces dispositions. Nuit totalement à l'attractivité du droit français parce que, outre l'imprévision qui franchement pas quelque chose qu'adorent les anglo-Saxons, quand on va leur dire en plus quand la prévision pourra être évoquée, un juge pourra remanier et refaire le contrat ça j'en suis certain le droit suisse passera avant le droit français, c'est donc contraire à l'objectif qui consiste à vouloir faire du droit français, un droit attractif, dernier point. Si nous prenons si nous contenues, de ses conséquences, je vous garantis que dans tous les contrats qui sont faits par des professionnels ont pas ceux qui se compte fait par des gens sans culture juridique mais tous ceux qui sont faits par des professionnels, ils écarteront. Les dispositions concernant la prévision vous viderait votre texte de son application, puisque c'est une disposition supplétive, je vous garantis, aucun avenir à ces dispositions, voilà les 4 raisons pour lesquelles je pense que nous ne devons pas nous ne devons pas. Agir pour changer la mission du juge dans notre système judiciaire, enfin, et parce que, dès l'origine, madame le ministre, vous avez bien vu que nous n'avons pas fait la réforme de la réforme que nous avons fait très peu d'amendements, même si la plupart de ceux que vous avez proposé moins est allez allez refuser, je vais quand même ouvrir une réflexion. Si un jour le juge pouvait être autorisée. à remodeler fiel contrat ça ne pourraient être conçues qu'avec l'accord des 2 parce que dès lors que c'est sous la demande d'un seul, vous avez déjà un désaccord, tels que le juge rendra une décision qui, de toute façon ne sera pas adopté dans un contrat qui s'exécutera entre 2 parties voilà toutes les raisons de pure pratique de, de, de cohésion Jéricho juridictionnel qui font que j'reste un notaire interprétation avec toutefois cette volonté. De vous dire que peut-être il y a du grain à moudre à la condition que le juge ne puisse être saisie à la demande des 2 parties. Merci, merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Collombat. Je crois qu'il faut savoir ce qu'on veut, ce qu'on veut introduire la notion d'imprévisibilité et en tenir compte ou pas. Moi je pense que c'est plutôt utile dans la mesure où c'est.

et sauf. Ce Président merci, juste pour le plaisir de de dialoguer avec monsieur le rapporteur, et avec vous, mesdames et messieurs les sénateurs, il me semble au contraire que revenir à la version initiale du texte, c'est finalement. Obtenir un texte assez équilibré, en effet, je ne partage pas votre sentiment lorsque vous dites finalement que la manière dont le texte est écrit en paralysera l'application car dites-vous, ce texte sera vidé de son effectivité, je ne le crois pas, je crois au contraire que c'est votre proposition, c'est-à-dire exiger un accord des 2 parties qui viderait le texte de sa substance, Monsieur le Sénateur, Colomba l'dit c'est-à-dire que il me semble au contraire que telle qu'il est rédigé le texte constitue une incitation puissante à négocier le fait qu'une seule des parties puissent demander finalement au juge de d'intervenir constitue un puissant moteur pour négocier et donc je pense que cette négociation d'ailleurs pouvant avoir lieu soit au moment de la conclusion du contrat, soit en cas d'inexécution liée à l'imprévision et donc il me semble qu'il y a là une riposte graduée, je crois d'ailleurs que si c'était un mécanisme aussi inefficace que vous le suggérez, monsieur sénateur ou en tout cas que vous imaginez des pays comme l'Allemagne ne l'aurait sans doute pas adoptée, or c'est bien le texte telle à peu près, telle que nous l'avons rédigée qui est adoptée en Allemagne. Madame Goulet demandé la parole. Oui, monsieur le président, le ministre, mes chers collègues, je voudrais simplement et soutient la position du rapporteur, probablement par nostalgie de Philippe Malaurie et de Malinvaud et du droit des contrats tels que telle que je l'ai appris mais mais aussi parce qu'on voit pas très bien le juge d'intervenir dans ces dans ce dans ce

Je veux dire Madame le Ministre, que déjà une taxe est un grand, grand progrès parce que l'imprévision. Préalablement, ne pouvait pas être évoquée, or dans le texte, le progrès que que je souligne que j'accepte, c'est le fait que le juge ce qui n'aurait jamais pu faire avant, va pouvoir prononcer la résolution et va pouvoir allouer des dommages et intérêts, ce qui n'aurait jamais pu faire moi ce que je conteste, c'est le pouvoir supplémentaire d'intervenir dans le contrat avec les responsabilités qui sont, qui sont afférentes à son intervention avec le désaccord d'une partie qui ne voudrait pas que le juge viennent viennent intervenir dans son contrat, raison pour laquelle je vous ai dit et ouvert la possibilité d'une discussion sur le fait que. Si le juge intervient à la demande des 2 parties, pourquoi ne consomme ferions-nous pas dans notre droit, un juge qui ressemblerait d'ailleurs fort un harnais. Mais en l'état, je maintiens ma construction intellectuelle, même si certains peuvent penser qu'elle est quelque peu boiteuses se confondent, moi je ne crois pas.

Nous passons. à l'amendement 30 2. Mais ça rapporte, il est purement rédactionnel, donc le gouvernement est favorable, merci Madame Lagarde Esso, qui est pour. qui est contre l'amendement est adopté je mais on voit l'article 13 qui est pour, qui est contre l'article 13 est adoptée Nous passons à l'article 9 et à l'amendement 6 rectifier bis présenté par Madame Mellow. Merci monsieur le président, l'article 221 nouveau du code civil, consacre le droit à l'exécution forcée en nature d'une obligation, ce droit est cependant limitée en cas d'impossibilité d'exécution ou de disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier, la proposition de la commission des lois de limiter la condition disproportion manifeste au cas où le débiteur et de bonne foi, va dans le bon sens, cette notion disproportion manifeste devrait cependant être encore plus strictement. Encadrés, c'est pourquoi le voile amendement propose d'insérer un après les mots disproportion manifeste, les mots et déraisonnable. Merci Madame Mellow quel est l'avis de la commission. peut-être redondantes avec celles de dispo disproportion manifeste donc une petite. Querelle d'écriture d'un avis défavorable. Peut-être estimerait vous que cela ne vaut pas le coup que nous nous je posions sur cet amendement.

au monde, ce dernier amendement précisait que tous, tous ces amendements ta bon soutenir l'attractivité du droit français, bon l'attractivité de la place de Paris

répondu à chacun des amendements et d'avoir donné des arguments qui qui ne paraissent recevable. Merci, cher collègue, nous passons à l'amendement 20 présenté par le gouvernement. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, je voudrais moi aussi vous remercier, madame la sénatrice du travail que vous avez proposé, même si nous n'avons pas suivi vos propositions, c'est vrai que la question du de l'interactivité de notre droit est tout à fait essentiel et je partage le gouvernement partage cet objectif quant à l'amendement dont je vous parle maintenant, il a pour objet de rétablir l'article 1221 de l'ordonnance dans sa rédaction initiale. Ce texte introduit en effet une modification importante du droit positif par rapport à l'ancien article 1142 du code civil qui posait le principe selon lequel l'inexécution des obligations de faire se résout en dommages et intérêts, l'article 1221 donc dans sa rédaction consacrent le principe inverse du droit à l'exécution forcée en nature du créancier d'une obligation toutefois comme tout droit dont l'exercice est susceptible de dégénérer en abus le droit exécution forcée doit connaître des limites, outre l'impossibilité d'exécuter l'article 1221 prévoit donc une exception au droit du créancier, l'exécution forcée en nature et détaille les conditions dans lesquelles l'exercice de ce droit serait constitutif d'un abus ainsi ne peuvent donner lieu à exécution forcée en nature, les cas dans lesquels il existe une disproportion manifeste entre le coût de cette exécution forcée pour le débiteur et son intérêt pour le créancier cette exception vise ainsi à mettre fin aux hypothèses d'abus qui ont pu être observées dans la jurisprudence, ce sont les cas par exemple de la construction d'une maison d'une hauteur inférieure de 33 centimètres ont pignon de celle d'une piscine dans l'escalier d'accès compte une marche de moins que prévu, que la Cour de cassation a eu à connaître et dans lesquels elle a ordonné l'exécution forcée en nature sans intérêt pour le créancier mais qui impliquait la destruction totale, puis la reconstruction de l'ouvrage à la charge du débiteur. L'objectif du texte et donc de mettre fin à de telles situations, il s'agit d'une déclinaison de l'abus de droit formulées de façon plus précise pour encadrer l'appréciation du juge et offrir une sécurité juridique accrue. La Commission, monsieur le rapporteur a proposé d'ajouter que l'application de ce texte est soumise à la bonne foi du débiteur, cette précision ne nous apparaît pas nécessairement utile et ce pour plusieurs raisons tout d'abord la bonne foi est déjà prévue à titre général à l'article 1104 nous l'avons déjà dit tout à l'heure, elle est un devoir des parties durant toute la vie du contrat et fonde tant techniquement que, philosophiquement, l'ensemble même de l'ordonnance de plus, la mauvaise foi éventuelle du débiteur et déjà sanctionné puisqu'il y a engagé par ailleurs sa responsabilité au-delà du dommage prévisible normalement seul réparable en matière contractuelle, conformément à l'article 1231 en outre l'exigence de bonne foi, s'applique tant aux débiteurs qu'aux créanciers, particulièrement dans l'usage que celui-ci fait des sanctions de l'inexécution prononcé à l'article 1217 la précision devrait donc être dans tous les textes relatifs aux parties au contrat tant pour le débiteur que le créancier et impliquerait de distinguer les textes pour lesquels pour l'application desquelles la mauvaise foi de la partie concernée serait indifférente à l'instar de l'article 1218 sur la force majeure, par exemple, et cela ne nous semble pas souhaitables : je vous demande par conséquent de bien vouloir mesdames et messieurs les sénateurs

lors de l'établissement de son texte, la commission a souhaité préciser que les séparations à l'exécution forcée en nature liés à la disproportion entre son coût pour le débiteur et son intérêt pour le créancier ne jouerait qu'en faveur du débiteur de bonne foi, pourquoi, parce que cette précision visait à éviter que cette exception ne constitue une incitation pour le débiteur existe c'est Sonobe légation de manière imparfaite, toutes les fois où le gain attendu de cette inexécution serait supérieur dommages intérêts qui pourraient être amenés à verser, il vise donc empêcher le débiteur soit de profiter de ce qui a été appelé dénommé pendant les auditions, une faute lucrative, voilà la raison pour laquelle nous avons ajouté le terme bonne foi cela dit n'pas été insensible à à à vos arguments, et en particulier à celui que j'évoquais tout à l'heure, à savoir. La bonne foi est un événement quasiment supérieur une auréole au-dessus du du texte, et c'est la raison pour laquelle j'en resterai à mon mandat de la commission, c'est-à-dire le mettre un avis défavorable mais que pour autant lors de la navette la discussion semble ouverte. Merci, monsieur le rapporteur, je vais mettre aux voix l'amendement du gouvernement qui a recueilli un avis défavorable de la commission, y a-t-il des explications de vote, je n'en vois pas qui est pour.

Il s'agit de donc de cette disposition qui permet à un créancier d'accepter une exécution non conforme, en en en contrepartie, donc d'une réduction de prix, l'objet de ces ces amendements, c'est à quelles conditions

l'article 1223 introduit dans le code civil, une nouvelle sanction à disposition du créancier. C'est d'une obligation mal exécuté, ce dernier peut, en effet, dans certaines circonstances se satisfaire d'une exécution même imparfaite de la prestation si le prix est proportionnellement réduits, le client pourra ainsi accepter la livraison de marchandises d'une marque différente de celle qu'il avait commandé ou promoteur se satisfaire de travaux réalisés avec des matériaux différents de ceux promis par l'entreprise, si le prix réduit néanmoins en pratique si le créancier a déjà payé le prix, il devra demander aux débiteurs remboursement d'une partie du prix et si ce dernier refuse, il n'aura d'autre choix que de saisir le juge, qui pourra prononcer la réduction judiciaire du prix. Ce n'est que si le créancier n'a pas encore payé qu'il pourra unilatéralement décider d'une réduction du prix il n'effectuera alors en effet qu'un paiement partiel que le débiteur, bien entendu, pourra toujours contester en justice s'il estime que cette réduction du prix et injustifiée la rédaction adoptée par la commission ne permet pas, selon moi, de comprendre ce mécanisme en indiquant au 1er alinéa que le créancier décide une réduction du prix, le texte est trompeur car le créancier, s'il a déjà payé doit s'adresser à son débiteur

dans sa rédaction antérieure aux travaux de la commission des lois. Or, prévoir que le créancier de l'obligation accepte son exécution est parfaite, alors même qu'il n'a reçu aucune offre en ce sens du débiteur n'a pas en enfance vraiment de logique de plus à partir du moment où le créancier de l'obligation décide la réduction du prix, voire même si l'on reprend le terme sollicité, qui sollicite une réduction du prix auprès du débiteur, on peut tout à fait considérer qu'il a de fait accepté l'exécution imparfaite de l'obligation s'agissant ensuite du terme sollicité que le créancier de l'obligation sollicite la réduction du prix ou la décide, cela ne change absolument rien dans les effets de la démarche du sommes puisque nous sommes dans une hypothèse ou le créancier a déjà acquitté le prix, donc je m'explique. Avec la rédaction qui serait issu de l'adoption de ces amendements le créancier pourrait solliciter du débiteur de l'obligation un parfaitement exécuté une réduction du prix si le débiteur refuser le créancier seraient contraints de saisir le juge dans le texte adopté par la Commission le créancier pourrait décider de réduire le prix de manière unilatérale, mais puisqu'il a déjà payé le prix si le débiteur de l'obligation refusait de rembourser la partie indument perçues le créancier comme dans la 1ère hypothèse c'est retour au problème précédent contraints de saisir le juge en revanche la rédaction choisi par la commission a me semble-t-il, le mérite de la clarté, il permet d'éviter d'avoir une rédaction qui diffère complètement, selon que le créancier à payer ou non, le prix de l'obligation s'il a déjà payé, il ne peut que solliciter la réduction, alors que s'il n'a pas encore payé, il peut l'imposer, il n'y a aucune justification à établir une différence dans le pouvoir de réduire le prix à partir d'un critère pris déjà payé ou non, qui ne l'explique pas, et je l'expliquais remplacer le mot sollicité par décider dans la 1ère dans la prairie, peut-être ne change absolument pas les effets de la procédure, enfin, alors même que le créancier subit une mauvaise exécution de l'obligation par le débiteur, il devrait le solliciter pour qu'il accepte de bien vouloir réduire le prix il y a là cette fois un véritable déséquilibre en faveur de la partie au contrat qui n'exécute pas correctement Sun obligation, c'est la raison pour laquelle la commission des lois, émis un avis défavorable à ces 2 arguments identiques. Merci, monsieur le rapporteur, je vais passer aux voix les 2 amendements identiques, il y a-t-il des explications de vote, je n'en vois pas qui est pour. Les 2 amendements identiques, ils ne sont pas adoptées. Je mets, on voit l'article 9 qui est pour. Qui est contre l'article 9 est adopté, nous passons à l'article 10 et un amendement 22, défendue par le gouvernement, madame Lagarde est sauf. sauf. Ce président, mesdames et messieurs les sénateurs, voici un amendement pour lequel je vais solliciter. Vos suffrages mais bien entendu vous déciderez alors l'article 1304 4. Consacrent la règle selon laquelle la partie dans l'intérêt de laquelle une condition a été stipulé au contrat peut renoncer tant que cette condition n'est pas réalisée, il est par exemple possible pour l'acquéreur d'un immeuble de renoncer à la condition suspensive d'obtention du prêt tant qu'il ne l'a pas obtenu la vente devient alors pu récente, à contrario, il n'est plus possible de renoncer après l'accomplissement de la condition et après la défaillance de celle-ci, cette solution est logique encadre fut de près par exemple le contrat est automatiquement anéanti, il ne peut donc renaître sans un nouvel accord des parties cette lecture est conforté par les termes du rapport au président de la République, force est de constater, toutefois, que l'interprétation du texte a été discuté par les praticiens je partage donc le souhait de la commission d'expliciter le sens du texte pour autant, le texte adopté par la commission me semble incomplet et ne reprend pas la règle selon laquelle la renonciation est possible avant l'accomplissement de la condition, je vous propose donc de rendre le texte plus clair en visant tant l'hypothèse de la réalisation de la condition, j'obtiens mon prêt par exemple que l'hypothèse de la défaillance de la condition, la banque refuse après la renonciation à la condition peut intervenir avant ces événements mais plus après. Pourtant même regarder sous cet amendement dont vise à modifier l'article 1384 du code civil pour prévoir que le bénéficiaire d'une condition suspensive ne peut plus y renoncer dès lors que cette condition est accompli ou des faits, la précision selon laquelle le bénéficiaire d'une condition suspensive puis renoncer tant la condition n'est pas accompli n'a pas d'intérêt, en effet, une fois que la condition est accompli que le bénéficiaire renonce ou pas les faits elle-même l'obligation est pure et simple, en revanche, le bénéficiaire doit pouvoir renoncer à la condition suspensive avant son accomplissement, ce qui est tout à fait possible grâce à la rédaction issue des travaux de la commission des lois, puisque le bénéficiaire peut y renoncer tant qu'elle n'est pas d'effet tant qu'il n'est pas défaillir, ça veut bien dire a contrario que le bénéficiaire peut renoncer. à la condition, tant qu'elle n'est pas accompli, voire même après son accomplissement, bien que cela se passe en effet comme je viens de l'expliquer la précision apportée par cet amendement m'apparaît inutile mais comme elle n'entraîne pas non plus une modification ou un bouleversement ou une interprétation radicalement différent de ce que je viens de dire si le gouvernement et tient vraiment la commission ne s'opposera pas à Hassan adoption c'est donc dire que la Commission va donner un avis de sagesse avec beaucoup de réserve, mais que, malgré ses réserves, je voterai votre amendement. Merci, monsieur le rapporteur, je vais donc mettre aux voix cet amendement qui a recueilli un avis de sagesse de la commission sagesse favorable. Qui est pour cet amendement qui est contre l'amendement est adopté je mais on voit l'article 10 qui est pour. Qui est contre l'article 10 est adopté, nous passons à l'article 11 et à l'amendement 23 défendue par Madame Lagarde. il s'agit ici de supprimer l'exigence décrit à peine de nullité pour la cession de dettes alors vous le savez la cession de dette permet à un débiteur de se libérer d'une dette en donnant à son créancier, un autre débiteur l'acquéreur d'un immeuble peut avoir intérêt à prendre en charge la dette d'emprunt de son vendeur, par exemple dans des relations d'affaires, il se peut également qu'une entreprise cette sa dette envers un fournisseur à une entreprise cliente débitrice à son égard. L'ordonnance a consacré, organiser la cession de dettes pour répondre aux besoins des praticiens et exigé qu'une telle situation se fasse nécessairement par écrit, à peine de de nullité de l'acte est-il nécessaire, il me semble que non, le principe en droit français, hé bien, en effet, celui du consensuel isthme les praticiens ne se ne sollicite pas : c'est écrit là c'est. Sur iTélé juridique ne l'exige pas les règles du droit de la preuve s'appliqueront le cas échéant en cas de contentieux les instruments concurrents tels que la délégation ne sont d'ailleurs pas soumis a écrit à peine de nullité, je vous invite donc, Mesdames et messieurs les sénateurs, à supprimer cette exigence.

est imposée par les dispositions du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance pour la cession de créances et la cession de contrat, il n'était pas exigé pour la cession de dettes, la commission des lois tout simplement souhaité harmoniser le formalisme qui s'attache à ses 3 types de scission, estimant qu'il n'y avait aucune justification, a exigé un écrit pour les 2 premières et pas pour la 3ème, pour cette raison, est défavorable à cet amendement qui supprime l'exigence d'un écrit pour les cessions sur le je dois dire que si ma mémoire me fait défaut, mais pendant les auditions, tous ceux qui se sont attachés à à l'article 11 ont, en règle générale, souhaité qu'il n'y a pas d'écrits pour les 3. Mais à aucun moment il n'ont accepté qu'il y a un écrit pour les 2 et pas pour la 3ème, donc c'est uniquement dans le cadre de l'harmonisation du droit. Que la commission a ajouté ce point et la raison qui fait que et la et demi un demi défavorable qu'elle maintient. Merci, monsieur le rapporteur, mais aux voix l'amendement qui a recueilli un avis défavorable de la commission. Pas d'explication de vote qui est pour. L'amendement 23 n'est pas adopté. Je maison voir l'article 11 qui est pour. Qui est contre l'article 11 est adoptée je mais on voit l'article 12 même vote. Même votre l'article 12 est adopté, nous passons à l'article 13 avec. Une parole. De Madame Mazetier chers collègues. Merci, merci Monsieur le Président Madame Lamy, triste, je voudrais vous interroger sur sur une évolution récente des conséquences juridiques de l'article 1343 3 du code civil article qui prévoit donc le paiement d'un contrat entre 2 entreprises éventuellement française qui peut s'effectuer dans une monnaie autre que l'Euro s'il s'agit d'une opération à caractère international ou d'un jugement étrangers dès lors aujourd'hui si le paiement se fait en dollars s'ouvre un risque juridique majeur pour nos entreprises ce que je voudrais souligner en effet aujourd'hui une transaction effectuée par des entités économiques non américaines et en dehors du territoire des États-Unis dès lors qu'elle est réalisée en dollar peut fonder la compétence extraterritoriale du droit américain et un rapport de l'Assemblée nationale sur l'extraterritorialité du droit l'année dernière, révèle qu'il suffit que ces opérations impliquent des ordres de paiement par le système international du Swift c'est-à-dire utilisent des chambres de compensation américaine pour ainsi assujettir aux lois américaines les transactions qui ont donné lieu à cette compensation cette projection extraterritorial du droit américain est motivée par la défense d'intérêts politiques et économiques, mais aujourd'hui, fort d'un pouvoir déterminant sur le fonctionnement des réseaux financiers des réseaux commerciaux et technologiques et à l'heure de la mondialisation, les États-Unis considère visiblement comme universelles leurs critères et leurs normes sur ce fondement, plusieurs entreprises européennes, notamment bancaires se sont vus dernièrement infliger des amendes colossales. je voudrais savoir, Madame la Ministre, comment vous appréhendez ces pratiques extérieures extraterritorial du droit américain, qui viennent et on peut le voir dans le cadre donc de l'application du droit des contrats éventuellement s'imposer aux entreprises et au droit français.

Le président merci oui je vais si vous le permettez, je répondrai à la question de madame la sénatrice peut-être enfin débat si vous y autoriser le temps que je réfléchisse en tout cas merci madame la sénatrice d'avoir posé cette question, j'en viens à l'amendement numéro 24 qui vise à préciser le texte sur le paiement aumône étrangère donc ce n'est pas sans lien avec la question vous avez posé. L'article 1343 tiré 3 a pour objet de codifier l'état du droit positif sur la faculté de payer une obligation en monnaie étrangère en effet aujourd'hui les règles applicables sont uniquement jurisprudentielle je souscris aux souhaits de monsieur le rapporteur, de préciser le texte afin de ne pas laisser penser que nous avons entendu restreindre les possibilités de payer un contrat en monnaie étrangère à cet égard l'expression opération à caractère international et plus proche de la jurisprudence que la référence à un contrat international qui peut-être entendu de manière plus restrictive l'amendement proposé par le gouvernement et donc ici purement rédactionnel, en effet, indiqué que le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie, s'il s'agit de procéder à une opération à caractère international viendrait restreindre la possibilité de la réception sur le sol national d'un paiement en une autre monnaie résultant d'une opération internationale, le gouvernement propose donc d'aligner la formulation sur celle qui prévaut dans l'article 1343 3 du code civil, dans sa version actuelle, en précisant que le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l'obligation ainsi libellé procède d'une opération à caractère international d'un jugement étrangers. Madame le ministre. Monsieur le rapporteur, la commission des lois avait ajusté sa rédaction pour tenir compte des observations du ministère de l'Économie et des finances que nous avons auditionnés le gouvernement souhaite apporter sans doute eu une amélioration à, à la rédaction qu'il a lui-même inspiré à l'avis favorable bien sûr. Merci, monsieur le rapporteur Madame Goulet pour l'explication de vote. Oui, Monsieur le Président, Madame le ministre japonais que c'est une c'est une disposition extrêmement importante en matière de de contrats internationaux,

dans un temps raisonnable cette mesure, c'est-à-dire le nombre de transactions qui auraient été faites en monnaie étrangère sur le sol français parce que ça pose aussi des problèmes d'adaptabilité et puis les problèmes de conversion et ça posera évidemment des problèmes et puis il y a un certain nombre de pays avec lesquels les transactions sont, ce ne sont pas faciles et qui pourrait stipuler des contrats en monnaie étrangère, je pense que c'est le prototype d'une excellente disposition mais qui va nécessiter une évaluation dans un délai dans un rapide comme nous avons toujours des disputes, des difficultés d'évaluation des dispositifs que nous mettons en place, je sollicite même gardé qu'avec le ministre de l'Économie et des Finances, on puisse, dans un délai de 18 mois ou 2 ans, évaluer l'impact de de cette mesure parce que je suis absolument persuadé qu'elle facilitera énormément et les transactions et l'attractivité de la place de Paris. Madame Goulet je mais au voile amendements plus d'explications de vote. Qui a recueilli donc un avis favorable de la commission qui est pour, qui est contre l'amendement est adopté je mais on voit l'article 13 qui est pour, qui est contre l'article 13 est adoptée je mais au voile article XIV même vote. Il est adopté, nous passons à l'article 15 avec un amendement 25 défendue par Madame Lagarde Merci monsieur le président, alors il s'agit ici de maintenir le texte à l'identique le texte donc régissant l'application dans le temps de l'ordonnance. Je comprends le souhait de la commission d'éviter que l'ordonnance ne s'applique à des contrats ou à des actes passés avant le 1er octobre 2016, date de son entrée en vigueur le gouvernement attaché à la sécurité des transactions partagent d'ailleurs ce souhait, c'est pourquoi l'article 9 de l'ordonnance prévoit expressément que ces dispositions ne s'applique qu'au contrat conclu à compter de cette date pour les actes juridiques antérieur, c'est le principe de survie de la loi ancienne qui s'impose l'ordonnance ne prévoit que 3 exceptions pour les 3 actions dites interrogatoire permettant de purger certaines situation juridique incertaine, aucune autre exception n'est prévue, le texte est donc sans ambiguïté aucune autre disposition même d'ordre public ne s'applique aux contrats antérieurs, la précision que la Commission souhaite adopter nous semble donc inutile, elle est d'autant plus inutile qu'elle ne répondra pas, me semble-t-il, à la préoccupation que vous exprimez monsieur le rapporteur, en effet, les décisions jurisprudentielles qui sont cités dans le rapport ne font pas application d'articles de l'ordonnance non encore entrée en vigueur, au motif qu'il serait d'ordre public ou qu'ils réagiraient les effets égo du contrat en réalité dans cette décision, la Cour de cassation interprète certaines règles anciennes non écrite à la lumière du droit nouveau issu de l'ordonnance sans pour autant appliquer directement celui-ci, je vous propose donc d'en rester aux règles simples fixés par les dispositions transitoires de l'ordonnance.

Engendré quelques discussions jurisprudentielle à la commission a donc voulu conforter la vie qui est entre nous, unanime, la question de l'application de l'ordonnance aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur est particulièrement débattu la position la plus simple, la plus largement partagée, qui est aussi celle retenue par la commission et de protéger l'attention des partis au moment où ils ont conclu le contrat en d'autres termes, la loi ancienne dans toute seule intégré doit se continuer à régir les contrats anciens, nous en sommes d'accord au nom de la liberté contractuelle de la sécurité juridique de la loyauté de la prévisibilité du droit au nom également de la protection constitutionnelle des contrats légalement conclus qui ne peuvent pas être remis en cause, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel que pour des motifs d'intérêt général, motif qu'on ne verrait pas ici plusieurs arrêts de la Cour de casser sur laissent penser qu'il voudrait bien appliquer de larges pans de la loi nouvelle aux contrats anciens, ce serait à mon sens une dénaturation et nous en sommes d'accord de l'intention du législateur et ce serait très discutable d'un point de vue constitutionnel, vous pensez que la rédaction nous évite ce risque, je ne crois pas, d'autre part, dans un arrêt du alors du 16 novembre 2016, mais nous verrons qui en a d'autres, la Cour de cassation a écarté un article rédigé de façon parfaitement similaire à l'article 9 de l'ordonnance prévoyant le maintien de la loi ancienne sauf exception expressément élite mythe hâtivement énumérées dans une affaire de bail d'habitation, c'est la preuve que la rédaction du gouvernement ne suffit pas d'autre part, dans 2 arrêts beaucoup plus récent et qui se font, application de l'ordonnance du 24 février du 21 septembre 2017 la cour interprète les règles anciennes du code civil, en matière de contrats au regard de la loi nouvelle en changeant en réalité leur portée, ce qui n'est pas satisfaisant, la rédaction de la commission, mais sans doute pas parfaite, mais il dit clairement l'intention du législateur, les contrats anciens doivent toujours être régis par la loi ancienne conformément à l'intention des parties qui sinon n'auraient peut-être pas, conclut nos travaux préparatoires ont une valeur qui doit absolument absolument éclairer le les magistrats, ce que je veux dire à amnistie c'est que nous poursuivons exactement le même objectif, nous ne sommes pas tout à fait d'accord sur le fait que sur la rédaction du texte, vous pensez que le texte suffit, moi je pense qu'il faut rajoute. C'est une garantie dans le même esprit que j'ai manifesté depuis le début de ces débats qui s'achève ce soir, et là, avec cet amendement, je pense que le gouvernement pourrait retirer cet amendement, estimant qu'en l'espèce, la protection supplémentaire qu'a apporté la Commission va tout à fait dans le sens de ses propres préoccupations. Merci, monsieur le rapporteur.

après le vote, alors qui est pour cet amendement. Qui a recueilli donc là l'avis défavorable de la commission qui est pour, qui est contre l'amendement 25 n'est pas adopté, je mais on voit l'article 15 qui est pour. Qui est contre l'article 15 est adopté. Madame la garde des Sceaux je vous passe la parole pour répondre à Madame Losier. Je vous remercie, Monsieur le Président, vraiment extrêmement brièvement à madame la sénatrice loisirs je comprends pleinement la préoccupation que vous avez émise, il est vrai que les juridictions Amérique. Ken retiennent largement leurs compétences en cas d'opération impliquant un paiement en dollars et il me semble cependant que le droit des contrats dont nous parlons ici n'a pas vraiment pour vocation à régler une telle difficulté la réforme dont nous discutons, je crois, rendra plus de le fait de soumettre au juge français des contrats internationaux, c'est d'ailleurs ce qui était mentionné dans le rapport. Canivet, dont l'un d'entre vous a fait mention tout à l'heure sur la question de l'attractivité de la place de Paris, mais vous avez raison et je crois que c'est une question question générale sur laquelle il convient de travailler à Madame, la sénatrice Goulet je voudrais dire que je suis bien sûr ouverte à une évaluation de la portée des dispositions de l'article 1343 3 du code civil, peut-être cette évaluation serait-elle pertinente à échéance de 18 mois ou de 2 ans pour bien mesurer l'impact de de ses éléments, je ne voudrais pas terminer mon propos sont remercier ici, la commission des lois, et remercier monsieur le rapporteur, le sénateur, vous avez compris le souci du gouvernement de stabiliser la situation situation juridique telle qu'elle était née de l'ordonnance du 10 février toutefois j'ai bien conscience que vos amendements étaient tous dans écrit dans une volonté constructive que je tiens ici à saluer et je tiens à vous remercier également Monsieur. Merci Merci madame la garde des Sceaux, je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi il y a-t-il des explications de vote. Je n'en vois pas. n'ai jamais aux voient l'ensemble du projet de loi ratifiant l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats du régime général et de la preuve des obligations. Qui est pour. Qui est contre. Le projet de loi est adopté. L'ordre du jour. Du mercredi 18 octobre 2017 à 14 heures 30 scrutin pour l'élection de 6 juges titulaires et de six juge suppléant à la Cour de justice de la République, conclusion de la commission mixte paritaire sur le projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, un autre à 14 heures 30, désignation de sénateurs, membres de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques écoutez les technologiques de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation de la délégation sénatoriale à la prospective de la délégation sénatoriale aux Outre- Mer et de la délégation sénatoriale aux entreprises, aux entreprises, à l'issue des conclusions de la commission mixte paritaire, prestation de serment des juges élus à la Cour de justice de la République, la séance est levée, je vous remercie.